La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 29 avril 2020 a été publié sur le site internet du Sénat.

Je rappelle également que, à l'exception de M. le Premier ministre pour sa déclaration, les orateurs s'exprimeront depuis leur place et que la tribune ne sera donc utilisée qu'une seule fois au cours de cette séance. Notre séance s'organisera en trois temps : après la déclaration du Gouvernement, la parole sera donnée à un orateur de chaque groupe, puis au Premier ministre pour leur répondre ; ensuite se déroulera une séquence de quinze questions-réponses ; enfin,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes à un moment critique. Lorsque, pour la première fois dans son histoire, notre pays se trouve confiné depuis plus de sept semaines, lorsque ses cafés, ses restaurants, ses universités, ses lycées et ses écoles, ses églises et ses temples, ses synagogues et ses mosquées, lorsque la très grande majorité de ses entreprises, la totalité de ses théâtres, de ses bibliothèques ou de ses librairies, et bien d'autres encore, sont fermés, vides de tout public, sans aucune activité, le moment est critique.

et sauver des malades, dont le nombre croissant a bien failli saturer les services de réanimation, le moment est critique. Lorsque des femmes et des hommes, en définitive peu nombreux,

nous sommes à un moment critique. Le moment est critique parce que, avec la France, c'est près de la moitié de l'humanité qui est confinée. Des nations entières sont comme désarçonnées, et même les plus grandes puissances paraissent désorientées.

Nous ne savons pas tout de ce virus- ce n'est d'ailleurs pas la moindre des leçons à tirer de cette crise sanitaire que de nous rappeler la masse infinie des choses que nous ne savons pas. Cela dit, il y a cinq mois, nous ne savions rien. La recherche a progressé à une vitesse qui force l'admiration, aussi bien sur la compréhension de la maladie que sur le séquençage du virus ou la mise au point des tests virologiques et sérologiques. La France est à la pointe des essais cliniques européens et mondiaux permettant de tester l'efficacité de traitements déjà utilisés pour d'autres pathologies. Avec la communauté internationale, nos chercheurs travaillent pour découvrir vaccins et traitements. Le virus nous fait violence, c'est indéniable. Il appelle réactivité et innovation, mais sans faire violence au temps de la science, de l'expérimentation et de la preuve. Ce temps demande de la rigueur, de la patience, de la chance aussi- j'espère que nous en aurons mais notre devoir est d'agir sans compter sur cette dernière, car des marges d'incertitudes, que nous n'avons jamais dissimulées ni sous-estimées, demeurent. Aucun pays au monde, aucun scientifique ne saurait aujourd'hui prédire l'été, l'automne, l'avenir qui nous attendent. Tel savant, affirmatif et catégorique, nous dit qu'il ne peut y avoir de deuxième vague et que l'été verra le virus disparaître ; tel autre, aussi savant et respecté, nous dit l'inverse. L'histoire dira sans doute lequel aura eu raison, mais je crains que nous n'ayons pas le temps d'attendre que l'histoire se fasse juge. Le moment est critique, parce que nous ne pouvons pas rester confinés. Le confinement a porté ses fruits grâce au civisme et à la discipline de nos concitoyens qui, dans leur immense majorité, ont compris la nécessité de respecter les règles exceptionnelles adoptées pour freiner l'épidémie. La propagation ralentit, le nombre de décès et d'entrées dans les services de réanimation baisse. J'ai déjà eu l'occasion de citer cette étude de l'École des hautes études en santé publique, qui estime que, pour le premier mois, le confinement aura permis d'épargner près de 62 000 vies. Si nos concitoyens n'avaient pas respecté le confinement, nos services de réanimation auraient de façon certaine été débordés : plus personne n'aurait pu y accéder et nos soignants auraient dû choisir entre les malades. C'est ce qui s'est passé dans certains pays, nous avons évité cette situation. Toutes les décisions que nous prenons restent guidées par cet impératif : protéger chaque vie humaine, ce qui implique très concrètement de veiller à ce que, à l'avenir, le nombre d'entrées dans les services de réanimation reste toujours inférieur aux capacités d'accueil. Pour atteindre cet objectif, chaque jour de confinement compte- il en reste six. Je mesure parfaitement l'impatience de nos concitoyens, qui souhaiteraient retrouver un quotidien normal, sans restriction et sans appréhension. Tout le monde aimerait renouer avec la vie d'avant, avec cette liberté inestimable de sortir pour travailler ou flâner, pour amener ses enfants au parc ou chez leurs grands-parents, pour s'offrir une soirée au restaurant, au théâtre ou entre amis, toutes choses qui n'ont rien d'accessoire, mais qui sont véritablement essentielles. Je mesure plus particulièrement combien le confinement pèse sur celles et ceux qui vivent dans des conditions précaires : ils sont au coeur de nos préoccupations. J'ai une pensée particulière pour ceux qui ont souffert de l'isolement en plus du confinement, notamment les personnes âgées seules chez elles ou coupées de leur famille dans les établissements d'hébergement pour personnes mais son coût social, humain et économique est colossal. Depuis le début du confinement, les passages aux urgences, les visites chez les généralistes ou les spécialistes, les vaccinations obligatoires pour les enfants, les campagnes de dépistage sont en chute libre, et c'est grave ! La lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les autres maladies, les autres dangers qui menacent nos concitoyens. Le Covid-19 est certes mais certains huis clos le sont aussi quand des violences, des négligences ou des renoncements s'exercent au sein de la famille. Le Covid-19 est toxique, mais le décrochage scolaire et social l'est tout autant. Nos enfants ont besoin d'être éduqués, cultivés, socialisés. Nos aînés et nos concitoyens les plus fragiles ont besoin d'être visités, accompagnés. Nos commerçants, nos artisans, nos industriels, nos entreprises et leurs salariés ont besoin de produire et de vendre. Leur angoisse n'est pas seulement de tomber malades, malades, c'est aussi parfois de mettre la clé sous la porte, de perdre leurs moyens de subsistance et, pour certains, ce qui donne un sens à leur vie. Le confinement crée, voire aggrave les difficultés que rencontrent certaines familles, certains secteurs, certains territoires. Depuis quelques jours, des tensions sont perceptibles dans certains quartiers sensibles, notamment la nuit. Nos policiers nationaux et municipaux, nos gendarmes font face à des actions parfois violentes, à des guets-apens. Nous imaginons tous la lassitude de nos forces de l'ordre et de nos concitoyens qui habitent dans des quartiers difficiles. Leur sentiment d'être assignés à résidence s'aggrave encore depuis sept semaines. Au-delà de ces violences sporadiques, le confinement déchire notre tissu social. Dès le début, les associations de lutte contre la pauvreté nous ont d'ailleurs alertés sur la hausse des dépenses auxquelles certaines familles étaient confrontées. que possible de nouveaux filets de sécurité : je pense à la prolongation automatique du versement des prestations sociales, à la prolongation de la trêve hivernale ou à l'ouverture de plus de 21 000 places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. Je pense au lancement d'un plan d'aide alimentaire d'urgence, distribuée notamment sous forme de tickets services. J'ai aussi annoncé qu'une aide exceptionnelle de solidarité serait automatiquement versée, le 15 mai, à 4 millions de familles pauvres et modestes

J'annonce aujourd'hui une aide pour les jeunes précaires ou modestes de moins de 25 ans. En raison du confinement, les restaurants universitaires ont fermé. Beaucoup de jeunes ont perdu les emplois dont ils ont besoin pour se nourrir et payer leur loyer. Certains jeunes se sont retrouvés dans une situation que je sais dramatique. Nous avons donc décidé de verser une aide de 200 euros à 800 000 d'entre eux. Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Elle sera versée à la mi-juin aux jeunes de moins de 25 ans précaires ou modestes, qui touchent l'APL. Nous avons mis en place tout un arsenal de mesures parmi les plus puissantes au monde pour soutenir notre économie. Je pense au chômage partiel, dont bénéficie plus d'un salarié du privé sur deux, aux prêts garantis par l'État pour soutenir la trésorerie des petites entreprises, entreprises, au fonds de solidarité pour les très petites entreprises et les travailleurs indépendants et, enfin, au report des charges fiscales et sociales. Il s'agit d'efforts considérables pour nos finances publiques, c'est-à-dire pour l'argent des Français, pour l'argent de la Nation nous sommes fiers qu'un grand pays comme la France sache les consentir. Pour autant, cette situation ne peut durer. Les fleurons de notre industrie sont menacés. L'aéronautique, l'automobile, l'électronique, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les start-up sont au bord de l'asphyxie. Tout ce qui participe au rayonnement de la France, comme le tourisme, les arts, la gastronomie, est à l'arrêt. Maintenir notre pays dans le confinement reviendrait à casser notre moteur économique, asphyxier nos poumons agricoles, à condamner notre attractivité, bref, à mettre en grand danger notre vie future, ainsi que la vie de nos enfants. Le moment est critique, parce que nous devons démontrer une forme de discipline collective pour apprendre à vivre avec le virus. Sans vaccin avant un bon moment, sans traitement à l'efficacité démontrée, sans immunité collective, c'est seulement par la prévention, la discipline, la rigueur des comportements individuels et collectifs que nous pourrons maîtriser l'épidémie. Un peu trop d'insouciance et de relâchement, et le risque d'une deuxième vague se préciserait. Un peu trop d'immobilisme et d'angoisse, et l'asphyxie collective serait inévitable. Tel est notre chemin de crête, d'autant plus délicat à aborder que les deux versants qu'il sépare sont des à-pics vertigineux. Sur ce chemin de crête, il nous faut avancer avec, dirais-je, une forme d'humilité combative. Le déconfinement aura lieu, pas à pas, avec des marches que nous espérons franchir toutes les trois semaines. Et quand je dis « nous espérons », cela signifie que nous pourrons rester parfois plus longtemps que prévu sur une même marche ou redescendre une marche si nécessaire. Pour y parvenir, notre stratégie est fondée sur trois principes : la progressivité, la territorialité, la réversibilité. Tous nos territoires ne progresseront pas au même rythme. Certaines régions, nous le savons tous, ont été frappées les premières et de plein fouet, comme le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Corse, la Bourgogne-Franche-Comté. À l'inverse, grâce au confinement national, de nombreux départements ont été épargnés. Le bon sens invite à ce que le rythme et les modalités du déconfinement s'adaptent aux spécificités de chaque territoire. Nos exigences en matière de santé publique et de reprise économique ont évidemment vocation à demeurer nationales, mais de nombreuses clés du déconfinement se trouvent sur le terrain entre les mains des acteurs locaux, notamment les maires et les préfets. C'est pourquoi j'ai engagé, avec les associations d'élus régionaux, départementaux et municipaux une concertation, que je crois étroite et que j'espère fructueuse. Depuis le 28 avril, nous avons progressé. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ici l'importance de ce travail collectif, mené au plus près des décideurs locaux. L'effort de discernement qui nous incombe doit être collectif autant qu'individuel, car il concerne nos institutions dans leur ensemble et chacun à son niveau : chaque famille, chaque personne âgée ou fragile, chaque travailleur, chaque élu, chaque fonctionnaire doit y concourir en conscience et en responsabilité. Ni les décisions de la puissance publique ni l'engagement du corps médical ne suffiront à vaincre l'épidémie s'ils ne sont appuyés par l'engagement civique et responsable de chacun. Il s'agit d'un moment critique, donc, d'un moment crucial même, au sens littéral du terme : nous sommes à la croisée des chemins. Devant l'Assemblée nationale, j'ai présenté les trois mots d'ordre qui président à notre stratégie de déconfinement : protéger, tester, isoler. S'agissant de la protection des Français, il faut le dire et le redire, les gestes barrières que sont la distanciation physique et le lavage des mains restent l'alpha et l'oméga de la sécurité. Avec ou sans masque, ils sont indispensables. Sur les recommandations des médecins, et dans la perspective du déconfinement, le Gouvernement a également décidé de recommander le port du masque, étant bien entendu que le masque ne vient pas en substitut, mais bien en complément des gestes barrières. Dans certaines situations où l'on est confiné, par exemple dans les transports publics ou dans une salle de classe, nous avons même décidé de le rendre obligatoire, dès que l'on est en âge de le porter. Nos concitoyens continuent à se demander s'il y aura, le 11 mai, des masques pour ceux qui le souhaitent. Pour beaucoup, l'angoisse d'une dépense supplémentaire est réelle. L'État, les collectivités territoriales, les entreprises travaillent main dans la main pour que les masques soient accessibles à tous sur tout le territoire à partir du 11 mai. Je remercie tous ceux qui ont pris des initiatives et qui se sont retroussé les manches. J'aimerais répondre au malentendu qui a échauffé ce week-end quelques esprits peut-être en mal de polémiques. Je dois dire que je peine à comprendre quel intérêt aurait eu la grande distribution à cacher des stocks de masques au lieu de les vendre en temps de pénurie. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de stocks cachés. Il y a des commandes massives et il faut un certain temps avant qu'elles ne se concrétisent en millions de masques disponibles pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour tous ceux qui pensent qu'il suffit de commander des masques pour les obtenir, j'ai un long historique dont je peux faire état. Mais ce qui compte pour l'instant, c'est que le 11 mai, chacun puisse se procurer des masques dans les commerces situés près de chez lui. Nous avons écouté les associations d'élus et resterons extrêmement attentifs à toutes les remontées du terrain. L'État et les collectivités locales assureront la protection de leur personnel. L'État financera 50 % des masques grand public que sont en train de se procurer les collectivités locales. À leur demande, j'ai décidé de prendre en charge, de façon rétroactive, une partie du coût de ces achats pour les commandes passées à compter du 13 avril dernier. J'ai appelé les collectivités qui en ont les moyens à faire preuve de solidarité envers les communes qui les entourent ou les plus petites collectivités. L'État réservera en outre une enveloppe hebdomadaire de 5 millions de masques grand public pour les plus vulnérables de nos concitoyens

Par ailleurs, les régions et l'État vont accroître leur soutien aux très petites entreprises et aux travailleurs indépendants, au-delà des initiatives déjà prises par certaines branches ou organisations professionnelles. Une plateforme de e-commerce vient d'être mise en place par La Poste, dont je tiens ici à saluer la mobilisation à nos côtés. le succès du déconfinement repose sur notre capacité à tester et à isoler les personnes atteintes du Covid-19. Depuis la semaine dernière, les élus, les préfets, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) disposent des éléments leur permettant de planifier la levée du confinement. C'est à l'échelle de chaque département que se déploiera cette chaîne formée de trois maillons, puisqu'elle commencera avec les tests, se poursuivra avec le traçage des éventuelles contaminations et s'achèvera, le cas échéant, par l'isolement des personnes contaminées. Les tests virologiques sont le fer de lance de notre stratégie de dépistage. Nous voulons, nous devons tester tous ceux qui présenteront des symptômes similaires à ceux du Covid-19, d'une part, et ceux de leurs contacts présentant un risque élevé de contamination, qu'ils soient symptomatiques ou non, Quand nous avons établi les modalités du déconfinement, le conseil scientifique nous indiquait que les modèles épidémiologiques prévoyaient entre 1 000 et 3 000 nouveaux cas par jour à partir du 11 mai. À chaque nouveau cas correspondra en moyenne le test d'au moins 20 à 25 personnes ayant croisé, dans les jours précédents, l'individu testé positif.

les laboratoires de recherche, les laboratoires vétérinaires sont mobilisés pour que ces tests soient accessibles à compter du 11 mai sur tous nos territoires. L'assurance maladie les prendra en charge à 100 %. J'aimerais toutefois insister sur un point : les prévisions épidémiologiques du conseil scientifique ont été formulées sous la condition d'un strict respect du confinement jusqu'au 11 mai. Quand on modélise, on doit partir d'un certain nombre d'hypothèses. L'hypothèse que nous avons retenue, c'est que le confinement resterait strictement observé jusqu'au 11 mai. En cas de relâchement- je ne le souhaite pas, mais il peut avoir lieu -, le nombre de nouveaux malades pourrait être bien supérieur aux prévisions qui ont fondé nos modèles, ce qui compromettrait la réussite de toute la stratégie que je viens d'exposer. Il est donc essentiel, je le dis avec gravité, de respecter scrupuleusement le confinement jusqu'au 11 mai. J'ai bien entendu ceux qui nous reprochent, ceux qui reprochent au Gouvernement de dire que, si les conditions n'étaient pas réunies, nous en tirerions les conséquences. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ose à peine imaginer ce qu'ils diraient si nous déconfinions, alors que les conditions initialement fixées ne se trouvaient pas réunies ! Pour réussir cette grande manoeuvre nationale de dépistage, de traçage et d'isolement, nous mobilisons plusieurs tours de contrôle. Les professionnels de santé libéraux, à commencer par les médecins généralistes, seront en première ligne pour identifier les malades et leur entourage familial immédiat. Les équipes de l'assurance maladie prendront ensuite le relais pour tracer les cas contacts. Enfin, si des apparaissaient, il reviendrait aux ARS et aux préfets de gérer ces cas, qui sont plus complexes encore. L'isolement des malades ou la mise en quatorzaine des cas contacts aura ensuite lieu à domicile, impliquant l'isolement de l'ensemble des membres du foyer.

propriétaires. Les ARS veilleront aussi au suivi sanitaire de ceux qui seront isolés dans ces structures particulières. cette chaîne de dépistage, de test et d'isolement dépendra du civisme de nos concitoyens. Nous ne vivons pas- fort heureusement, mesdames, messieurs les sénateurs ! -dans un régime policier. Pour cette nouvelle phase qui commence le 11 mai, l'assouplissement du confinement s'accompagne nécessairement d'un assouplissement des contrôles. s'agit donc d'un défi logistique, bien entendu, mais aussi d'un défi civique qu'il nous faut relever. Ce défi logistique nécessite une organisation qui impose de recourir à des instruments nouveaux. Dans le texte que le Sénat examinera dans quelques heures, une disposition permet aux équipes constituées pour remonter les chaînes de contamination de faire le travail, d'appeler les cas contacts, de leur indiquer les lieux où se faire tester ou être isolé, de vérifier que les procédures ont bien été respectées. Sans le fichier permettant à ces brigades de fonctionner, nous n'avons aucune chance de remonter de façon systématique les chaînes de contamination et, donc, de maîtriser la propagation de l'épidémie. Le défi de l'organisation et du civisme concerne également la réouverture des écoles et des crèches. Là encore, nous sommes attentifs à toutes les complexités de mise en oeuvre, ouverts à toutes les propositions, conscients des innombrables spécificités d'un territoire à l'autre ou d'une classe à l'autre. Mais, avant de poser ces difficultés, nous devons rappeler que la fermeture des écoles est, à l'évidence, une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents. Celles et ceux qui n'ont pas accès à des livres ou à internet, celles et ceux qui n'ont pas toujours accès à une alimentation correcte, celles et ceux qui n'ont pas un espace à eux pour respirer et qui se sentent livrés à eux-mêmes doivent pouvoir retourner à l'école. Cinq mois de décrochage scolaire pour des dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement. Le confinement pose beaucoup de bombes à retardement de toutes natures, aussi bien sociale qu'économique ou géopolitique. Il me semble que celle-ci n'est pas la moins dangereuse. La réouverture des écoles nous semble donc une priorité pédagogique, sociale, républicaine, qu'il faut évidemment concilier avec nos impératifs sanitaires. Les préfets, les recteurs, les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale y travaillent sans relâche. Les effectifs ne devront pas dépasser quinze élèves par classe pour favoriser le respect des gestes barrières. Du gel hydroalcoolique sera distribué et la vie scolaire devra être aménagée pour assurer le contrôle des flux d'entrée, ou encore la restauration scolaire quand elle reprendra. En ce qui concerne le calendrier, comme je l'ai indiqué, nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et des écoles élémentaires à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat.

Nous déciderons à la fin du mois de mai si nous pouvons rouvrir les lycées, en commençant par les lycées professionnels début juin. Comme je l'ai également déjà dit, nous fournirons des masques aux personnels de l'éducation nationale et aux collégiens. Pour ces derniers, le masque sera obligatoire quand les règles de distanciation sociale risquent de ne pas être respectées. Pour les élèves des classes élémentaires, le port du masque n'est pas recommandé ; il est même proscrit pour les enfants de maternelle. Le 11 mai, tous les enfants et tous les adolescents ne retourneront pas physiquement à l'école. La situation ne sera pas identique dans toutes les écoles de toutes les communes, dans toutes les classes d'un même niveau. À la vérité, l'était-elle avant le confinement ? On pourrait en débattre ... Mais je suis intimement convaincu que, là où la réouverture peut avoir lieu, elle doit avoir lieu, si possible pour les enfants qui en ont le plus besoin. Je sais bien, mesdames, messieurs les sénateurs, nous savons bien que tous les enfants en ont besoin, mais il est un fait que certains en ont probablement encore plus besoin. Il est certain que les directeurs d'école, les professeurs, les services de l'éducation nationale, les maires peuvent faire en sorte que ceux-ci, et d'autres, puissent reprendre le chemin de l'école. Ne disons pas d'emblée que, parce que la reprise ne serait pas possible partout, elle ne devrait avoir lieu nulle part. Chaque retour à l'école sera une bonne nouvelle. J'en appelle donc, là encore, au discernement de chacun- familles, équipes pédagogiques, rectorats -pour que les groupes de quinze élèves soient formés de jeunes issus des familles qui en ont le plus besoin. Les autres continueront à travailler et n'interrompront pas leur scolarité : ils pourront le faire chez eux ou dans les locaux scolaires ou périscolaires mis à la disposition des collectivités, lorsque la disposition des locaux s'y prête et lorsque cela est possible. Les mêmes contraintes et, donc, le même civisme s'imposent aux crèches. Les enfants seront accueillis par groupes de dix. Je sais que les professionnels de la petite enfance mènent un travail remarquable et qu'ils décideront, au cas par cas, quelles sont les familles prioritaires. Je remercie très sincèrement celles et ceux qui s'occupent des enfants dans ces circonstances éprouvantes. S'agissant des entreprises, le télétravail doit se poursuivre après le 11 mai pour limiter le recours aux transports en commun et favoriser la distanciation physique. Quand le télétravail est impossible, il faut encourager la pratique des horaires décalés et limiter la proximité des salariés dans un même espace de travail. C'est facile à dire, mais c'est évidemment difficile à mettre en oeuvre, surtout dans les grandes agglomérations où l'organisation de rythmes différents peut s'avérer délicate. Il n'empêche que les collectivités territoriales, les autorités organisatrices de transport, les responsables et les représentants des entreprises peuvent, me semble-t-il, tenter de s'entendre pour améliorer la donne et la situation. Sur la question des transports, les inquiétudes sont grandes. Pour les transports interrégionaux et interdépartementaux, c'est-à-dire pour effectuer des trajets de plus de 100 kilomètres, les déplacements devront être réduits au motif impératif qu'ils soient familiaux et professionnels. Lorsque ces déplacements auront lieu en train, il sera assez facile, par un système de réservation obligatoire, de limiter l'accès aux voitures à la moitié de la capacité normale et de diminuer, ce faisant, la densité et la proximité des voyageurs. L'exercice sera, bien entendu, beaucoup plus compliqué dans les transports en commun, singulièrement dans les zones les plus denses comme dans les grandes agglomérations régionales. Je pense, notamment, à celles qui sont dotées d'un métro. évoqué l'éthique de responsabilité et la nécessité pour chacun de se montrer à la hauteur du moment que nous vivons, à l'instar des personnels hospitaliers, qui se sont littéralement surpassés ces dernières semaines pour trouver de la place pour tous les malades et nous permettre de surmonter la première vague de l'épidémie. Dimanche, c'est d'abord par la presse que j'ai pris connaissance d'une lettre adressée au Premier ministre par des responsables d'entreprises de transport- publics, pour beaucoup d'ailleurs -exprimant leur crainte de ne pas savoir organiser les services publics dont ils ont la charge, dans les conditions que le Gouvernement et le Parlement jugent nécessaires à la réussite du déconfinement. Ne voulant voir dans ce procédé que le souhait de surmonter au mieux les difficultés qu'ils anticipent, j'ai demandé au secrétaire d'État chargé des transports d'intensifier encore ses échanges avec eux afin qu'ils trouvent les bonnes réponses aux questions complexes que soulève l'impératif d'une ouverture maîtrisée des transports publics à compter du 11 mai. Je ne doute pas qu'ils sachent y parvenir, animés par cet esprit de dévouement au bien public qui permet à tant de nos concitoyens de se surpasser dans leur tâche depuis l'arrivée du virus sur notre sol. La vie économique, mesdames, messieurs, doit reprendre impérativement et rapidement, avec des aménagements et de la bonne volonté. Les fédérations professionnelles et le ministère du travail ont réalisé des guides et des fiches métiers pour accompagner les réorganisations nécessaires au sein des entreprises. fiches soient aujourd'hui disponibles. Tous les secteurs en auront à disposition le 11 mai. Les partenaires sociaux jouent un rôle précieux pour que ces plans de réorganisation du travail respectent au mieux les gestes barrières. Je me suis entretenu jeudi dernier avec les syndicats de salariés et les représentants des employeurs pour que le dialogue social contribue à remettre la France au travail sans mettre en danger la santé des Français, ce qui implique aussi de continuer à accompagner les entreprises en difficulté. Le dispositif d'activité partielle, que nous avons mis en place, et qui est l'un des plus généreux d'Europe, restera en vigueur jusqu'au 1 juin. Nous l'adapterons ensuite progressivement selon l'évolution de l'épidémie. Le fonds de solidarité sera prolongé jusqu'à la fin du mois de mai, il sera même renforcé pour les très petites entreprises (TPE) qui ont fait l'objet de mesures de fermeture administrative. Le deuxième étage de ce fonds, qui donne droit à une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 euros, sera désormais accessible à tous les commerces qui ont été fermés, y compris s'ils n'ont pas de salariés, ce qui est souvent le cas pour les coiffeurs, les fleuristes ou les libraires. Les reports de charges fiscales et sociales resteront autorisés jusqu'à la fin du mois de mai. Nous sommes prêts à convertir ces reports en exonérations définitives de charges, non seulement pour les entreprises du secteur de la restauration et du tourisme, mais aussi pour toutes les TPE ayant fait l'objet de mesures de fermeture. Ces mesures exceptionnelles témoignent de notre détermination à soutenir toutes nos entreprises pour qu'elles puissent repartir le plus vite et le mieux possible. C'est aussi pour relancer notre moteur économique que nous avons décidé de rouvrir les commerces, les marchés de plein air, les halles couvertes. L'ensemble des associations d'élus le demandaient, nos concitoyens y sont favorables là encore, ils devront respecter strictement les règles de distanciation physique qui prévalent. Les préfets pourront refuser leur ouverture si ces règles ne sont pas respectées. Ils pourront également décider de ne pas laisser ouvrir au-delà des sections alimentaires les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés, qui attirent et brassent des populations bien au-delà des bassins de vie. Ce n'est pas de gaieté de coeur, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous avons choisi par précaution sanitaire de prolonger la fermeture des restaurants, des cafés, des cinémas, des théâtres, des manifestations sportives et culturelles, des plages, des lacs, des salles de fêtes. La situation sera réévaluée fin mai pour une décision effective au 2 juin. Le retour à la vie normale sera donc progressif et adapté à chaque territoire. Jeudi dernier, le ministre des solidarités et de la santé a présenté à nos concitoyens une carte de France tricolore. Chacun a pu ainsi savoir si son département était classé en zone rouge, verte ou orange au vu des critères définis avec les autorités sanitaires. Cette carte de France sera actualisée chaque jour, en toute transparence. Elle deviendra rapidement bicolore : nous avons classé pour l'instant en orange les zones qui étaient encore en évolution incertaine. Notre stratégie de lutte contre l'épidémie a été déclinée avec la plus grande vigilance dans nos outre-mer. Il en va de même pour notre stratégie nationale de déconfinement. Je suis très Je suis très attentif à ce que ces territoires disposent, comme l'Hexagone, des tests et des masques grand public, notamment dans les crèches, les écoles, les transports. La chaîne de vigilance, de suivi, de responsabilité, doit être partout aussi résistante grâce aux élus locaux et aux préfets. J'ai parlé de différenciation : outre-mer, la principale adaptation de la stratégie nationale porte sur le maintien des interdictions d'arriver dans ces territoires au-delà du 11 mai. Seules les personnes ayant des motifs familiaux ou professionnels impérieux, ou une obligation de santé, pourront se rendre outre-mer. Elles demeureront soumises à l'obligation de quatorzaine. Nous effectuerons un point début juin afin de voir s'il faut maintenir ces mesures très contraignantes, qui pèsent évidemment sur les capacités de fret. Je tiens néanmoins à indiquer que nous profiterons du déconfinement pour organiser le retour chez eux des étudiants ultramarins qui en ont exprimé le souhait dans le cadre du recensement qui vient de s'achever. Je dirai enfin un mot sur Mayotte où nous avons choisi de reporter le déconfinement. Mayotte vient de passer en phase 3. Le virus y circule activement. La prolongation du confinement est l'unique manière d'éviter la saturation d'un système hospitalier déjà très sollicité et fragile. Nous ferons un point le 14 mai pour envisager l'assouplissement du confinement, en particulier le retour à l'école primaire à partir du 18 mai. D'ici là, nous continuerons à renforcer les capacités sanitaires du territoire, ainsi que les actions pédagogiques et sociales que nous y menons, notamment en matière d'aide alimentaire. Je finirai, mesdames, messieurs les sénateurs, en évoquant trois emblèmes de ce que signifie, pour notre pays, « vivre » dans le sens le plus plein du terme : la vie culturelle, la vie cultuelle et les élections municipales. La liberté de créer, de se laisser bouleverser et habiter par des oeuvres d'art, le droit de voter et de se présenter à des élections, la liberté de culte sont parmi les libertés les plus sacrées que nos concitoyens exercent et revendiquent. Mais alors que l'appétit culturel des Français est comme décuplé par le confinement, le secteur culturel est l'un des plus frappés par la crise sanitaire. Cette dernière met au jour et accroît la vulnérabilité de milliers de professionnels et d'innombrables institutions. Il y a urgence pour la culture, le Gouvernement le sait et travaille à trouver des solutions. Dès le début du confinement, nous avons garanti l'accès des acteurs de la culture aux mesures d'urgence mises en place par le Gouvernement. Le secteur des arts et de la culture a pour l'instant bénéficié de 52 millions d'euros du fonds de solidarité. Par ailleurs, comme l'a annoncé le Président de la République la semaine dernière, les acteurs de la culture sont éligibles au plan de 8 milliards d'euros d'accompagnement des secteurs particulièrement impactés, comme le tourisme et les cafés ou restaurants. Les difficultés mises au jour, comme la question du chômage partiel pour les intermittents, l'accès des artistes auteurs au fonds de solidarité ou l'accès des entreprises aux prêts garantis par l'État, seront réglées dans les prochains jours. Les ministères de la culture, du travail et de l'économie s'y emploient. Le Gouvernement a également mis en place des mesures d'urgence spécifiques pour les acteurs culturels. Certaines situations sont dramatiques, et il faut continuer à soutenir et à protéger la création. Le Président de la République annoncera de nouvelles décisions mercredi. Nous avons d'ores et déjà décidé de rouvrir de premiers lieux culturels à partir du 11 mai, dans le respect des exigences sanitaires. Ce sera notamment le cas des lieux culturels de proximité, qui participent à la vie éducative de nos enfants- les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les monuments -, dont la fréquentation n'entraîne pas

Nous devrons attendre début juin, si la situation sanitaire le permet, pour rouvrir tous les lieux de spectacle, les salles de cinéma et les grands musées et monuments. Il conviendra alors d'examiner dans quelles conditions tous

de tous ceux qui contribuent au succès de ces manifestations d'importance. Nous aurions tous aimé que le festival d'Avignon, les Francofolies, les Eurockéennes, les Nuits de Fourvière aient lieu. Mais il n'est pas possible de concilier ces grands rendez-vous culturels avec les précautions sanitaires nécessaires à la gestion de l'épidémie. Notre priorité, c'est d'éviter l'irruption d'une deuxième vague. Le même état d'esprit nous anime en ce qui concerne la liberté de culte. J'entends le désarroi des croyants, privés de rassemblements et de célébrations, qui ne sont pas seulement une expression de leur appartenance religieuse, mais sont aussi l'une des sources vivantes de leur foi. Ils ont dû renoncer à beaucoup de ces rites qui marquent les grands moments de la vie. Je pense aux moments de fête autant qu'aux moments de deuil. Je comprends l'impatience des ministres du culte de toutes les confessions. Je leur demande instamment d'attendre, en conscience, pour que nous n'ayons pas à regretter une décision précipitée. Tout le monde reconnaîtra que les cérémonies et offices dans les églises, dans les synagogues, dans les temples ou dans les mosquées, et à plus forte raison les mariages, les baptêmes, les bar-mitsva, réunissent des proches et des moins proches, dans des lieux souvent confinés, avec une forme de brassage qui est profondément réjouissante en temps normal, mais infiniment périlleuse en temps de crise sanitaire. J'avais indiqué qu'il faudrait attendre le 2 juin pour que les offices et les prières ouvertes aux fidèles puissent de nouveau se tenir dans les lieux de culte. de culte ont fait des propositions, après s'être entendus, pour concilier le déroulement de leurs réunions avec les exigences de distanciation physique. Je sais, notamment, que la période du 29 mai au 1 juin correspond pour plusieurs cultes à des fêtes ou à des étapes importantes du calendrier religieux. C'est pourquoi, si la situation sanitaire ne se dégrade pas au cours des premières semaines de levée du confinement, le Gouvernement est prêt à étudier la possibilité que les offices religieux puissent reprendre à partir du 29 mai.

Dans les 30 000 communes qui ont élu un conseil municipal complet, beaucoup plaident pour une installation rapide des équipes qui disposent depuis le 15 mars de la légitimité du suffrage. C'est un enjeu démocratique puisque le scrutin est terminé C'est aussi un enjeu économique, car leurs administrés comptent, bien entendu, sur eux pour prendre des décisions en matière d'investissement. La loi du 23 mars 2020 a fixé le cadre dans lequel nous devons nous placer pour prendre les décisions essentielles que sont l'installation des conseils municipaux élus au premier tour et la possibilité de tenir le deuxième tour des élections. L'article 19 de cette loi dispose que Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l'état de l'épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant. Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre : « 1° Pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ; « 2° Pour les réunions des conseils communautaires. communautaires. » Rien n'impose, dans cet article, que le comité de scientifiques statue en une seule fois ou que le Gouvernement fasse un rapport unique sur ces questions. Autrement dit, le Gouvernement peut demander un avis au conseil scientifique sur la question de l'installation des conseils élus et des conseils communautaires sans attendre le 23 mai. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi ce matin le conseil scientifique sur ces deux questions- et sur ces deux questions-là uniquement. Sur la base de son avis, je remettrai au Parlement un rapport dans les plus brefs délais. Il s'agit de déterminer

Les dispositions de l'article 10 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui prévoient que chaque élu peut détenir deux procurations, au lieu d'une actuellement, et qui assouplissent les conditions de quorum, puisque seule la présence d'un tiers des membres est requise, permettront de concilier plus simplement le respect des conditions de sécurité sanitaire et le bon fonctionnement de la démocratie locale. S'agissant du deuxième tour, je crois qu'il importe d'attendre encore un peu. Je remettrai au Parlement, au plus tard le 23 mai, comme la loi me l'impose, le rapport qui déterminera si ce deuxième tour peut avoir lieu en juin. Dans le cas contraire, nous devrions décider collectivement, d'une part, de sa date et, d'autre part, des modalités de son report, report qui emporterait avec lui un certain nombre de conséquences que personne ici n'ignore. Le Gouvernement et moi-même consultons très régulièrement les associations d'élus et les groupes parlementaires, et nous continuerons à le faire, pour préparer cette échéance. Enfin, j'entends les réticences de certains maires et de certains chefs d'entreprise, qui craignent que leur responsabilité ne soit engagée. Le sujet de la responsabilité face aux Covid-19 n'est pas une petite question. J'aimerais donc m'y attarder un peu. Le régime de responsabilité pénale des décideurs vous est bien connu. Il est issu, en plus des dispositions anciennes du code pénal, de la loi dite « Fauchon » du 10 juillet 2000. Si ce régime n'a pas été modifié depuis près de vingt ans, c'est qu'il est juste, c'est-à-dire qu'il est à la fois précis dans son contenu et équilibré dans sa portée.

Chacun sait, en outre, que ces dispositions n'ont pas empêché des responsables publics de répondre- car être responsable, étymologiquement, c'est bien d'avoir à répondre -de leurs décisions. Il n'en reste pas moins que la question se pose et que les inquiétudes sont là. Il nous faut donc y répondre.

Bien entendu, le Sénat est parfaitement dans son rôle quand il accorde une attention particulière à la situation des élus locaux. Pour autant, un maire qui rouvre une crèche, un président d'intercommunalité qui organise les transports en commun, un préfet qui autorise la reprise d'un marché ou un chef d'entreprise qui redémarre un chantier ne sont pas dans des situations fondamentalement différentes. Il s'agit chaque fois de femmes et d'hommes qui ont la responsabilité d'autres femmes et à qui il incombe de prendre des décisions durant cette crise. Traitons-les de façon équitable. Deuxièmement, cette question mérite d'être traitée avec prudence, car nos concitoyens veulent que les maires agissent sans blocage. Mais ils ne veulent pas non plus que les décideurs- publics ou privés -s'exonèrent de leurs responsabilités. Je le redis, ce n'est en rien un hasard si les termes de la loi Fauchon n'ont pas bougé depuis vingt ans. Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont,

soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » Il me semble, mais il appartiendra au Parlement d'en décider, que nous devons préserver préciser la loi, rappeler la jurisprudence qui oblige le juge à tenir compte des moyens disponibles et de l'état des connaissances au moment où l'on a agi ou pas. Mais je suis nettement plus réservé Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, c'est ensemble que nous devons résoudre les problèmes, pas à pas. J'y suis disposé. Il appartiendra au Parlement de trancher la délicate question de savoir si ce sujet sérieux, ce sujet qui suscitera beaucoup d'attention, pas simplement de la part des décideurs, bien entendu, la part de l'ensemble de nos concitoyens, doit être traité à l'occasion d'un amendement ou d'un texte spécifique. J'ai la certitude que le Parlement dans son immense sagesse saura répondre à cette question délicate. Le 11 mai, mesdames, messieurs les sénateurs, ne sera pas le début de l'insouciance : ce sera le début de la reprise. Il faut nous y engager avec prudence et responsabilité. Pendant des siècles, quand survenait une épidémie, on se répétait le fameux que l'on peut traduire par « pars vite, loin et longtemps », que la tradition attribuait à Galien,

et pour nous moins que pour quiconque, de fuir, de nous dérober face à cette épidémie. Il est question de prendre de bonnes décisions qui engagent toute la collectivité, sans fuir le débat, en mettant le Parlement au coeur des enjeux. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous présenter notre stratégie nationale de déconfinement et à la soumettre à votre vote. Nous présenterons aussi cette semaine au Parlement une loi qui vise à proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet prochain et qui tend à autoriser la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'accompagnement du déconfinement. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous voulons, comme nos partenaires européens, traverser l'épreuve de cette épidémie dans le respect de nos valeurs. Nous voulons démontrer que la démocratie libérale et sociale est capable de faire face. Quand une démocratie comme la France est à la croisée des chemins et qu'il faut définir, puis emprunter, les voies les moins mauvaises, les moins périlleuses pour nos concitoyens, elle ne peut y parvenir qu'avec le soutien et l'apport d'élus représentant les Français, dans toute leur diversité et au plus près de nos territoires. Cette conviction sous-tend mon engagement politique, elle est un fil directeur de notre action. La réussite de ce déconfinement reposera sur l'adhésion de nos concitoyens, qui est un moteur infiniment plus puissant que la contrainte. Ce qui se joue avec ce déconfinement, c'est un acte de confiance collective- pas seulement un acte de confiance entre citoyens ou entre nous, dans cet hémicycle, mais

Les épidémies de l'ampleur de celle que nous traversons ne sont jamais anecdotiques dans l'histoire d'une civilisation. Elles peuvent conduire à l'affaiblissement, peut-être même à l'écroulement. Elles peuvent aussi amener à une forme de rénovation. Comme vous, je crois en mon pays. J'ai la conviction la plus inébranlable que nos institutions, nos talents, notre jeunesse sauront nous relever de cette crise avec un surcroît de force et de solidarité. Nous en

qui ont participé à l'effort de la Nation en matière sanitaire, mais aussi en matière économique. Cette situation dramatique et inédite, le Gouvernement- avec l'ensemble des Français -l'a affrontée, et continuera de l'affronter, avec responsabilité et pragmatisme. La décision de mettre en place des mesures de confinement a été prise avec sang-froid et lucidité. Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais un instant revenir sur les jugements hâtifs ou autres critiques contradictoires, qui ne me semblent pas être à la hauteur de la situation à laquelle nous sommes collectivement confrontés. Dans un réflexe pavlovien, certains critiquent avec autant de ferveur les mesures du déconfinement que celles du confinement, qu'ils avaient pourtant décriées à l'occasion de leur mise en oeuvre. Ils critiquent par avance toutes les mesures proposées, ils énoncent leurs certitudes sur l'avenir, alors qu'ils ont été bien incapables d'anticiper par le passé Le déconfinement, qui n'est pas la sortie du tunnel, doit être préparé avec toutes les inconnues propres à ce fléau sanitaire. La tâche est immense, et c'est la raison pour laquelle est organisé ce débat

nécessaire à bien des égards puisque, depuis le 17 mars, les Français sont confinés pour préserver leur santé, notre santé. Au cours des deux derniers mois, nous avons mesuré combien la liberté d'aller et de venir, celle d'interagir avec nos proches, notre famille, celle de tisser des liens avec nos semblables, est consubstantielle à notre condition. Afin de renouer avec cette part de nous-mêmes, le déconfinement est nécessaire. Il est également nécessaire, voire plus encore, car la crise économique et sociale, qui impacte notre pays comme tous les autres, aura des conséquences lourdes que chaque Français doit intégrer. Le redémarrage de notre économie est un préalable indispensable à la reconstruction de notre nation. Cette récession qui s'annonce menace en premier lieu les plus fragiles sur le plan économique. Elle pourrait être rapidement synonyme de régression sociale si rien n'avait été prévu.

Monsieur le Premier ministre, vous l'avez souligné, ce déconfinement est risqué. Il est risqué, parce qu'il dépend de facteurs inhérents à l'épidémie et parce que les décisions à prendre sont complexes, et délicates. Si votre gestion pragmatique de la situation sanitaire est à saluer, tâchons de reconnaître la part d'incertitude qui existe quant au devenir de cette maladie virale. Bien malins ceux qui, sur les réseaux sociaux ou autres plateaux de télévision, prétendent connaître l'évolution du Covid-19, sa date d'expiration et l'heure de sa disparition Toutes ces suppositions et supputations alimentent le registre du commentaire alors que nous devons collectivement nous retrouver dans celui de l'action. Monsieur le Premier ministre, ce déconfinement ne peut aboutir que s'il est entendu de façon claire et précise. Il ne peut aboutir que s'il est appliqué de manière progressive, et exercé avec civisme et rigueur par les Français. Dans le même temps, les craintes et inquiétudes légitimes de nos concitoyens doivent être entendues. C'est ce que vous faites quotidiennement avec l'ensemble des membres du Gouvernement. Il importe d'appliquer à la lettre la règle des quatre C : clarté, cohérence, cohésion et concertation. La clarté est l'axiome principal de la politique qui doit être menée : la clarté en matière sanitaire, par exemple. J'ai entendu la polémique sur les masques. Je ne voudrais pas qu'elle fasse oublier les milliards d'euros que toutes les mesures mises en oeuvre aussi bien dans le domaine économique et social que dans le domaine sanitaire. À ce titre, je tiens à saluer l'objectif de 700 000 tests par semaine, ainsi que la remontée d'informations permise par les brigades que vous avez récemment évoquées. La clarté, nous la devons également à nos élus, bien évidemment aux maires, qui font remonter leurs inquiétudes. Vous le savez, monsieur le Premier ministre, ceux-ci évoquent notamment leur crainte de voir leur responsabilité pénale engagée à l'occasion de la réouverture des écoles. Vous venez d'y répondre par avance. Je sais bien que, aujourd'hui, le droit les protège- la loi Fauchon, en l'occurrence, comme vous l'avez rappelé. Encore faut-il qu'elle soit bien précisée pour que chacun soit rassuré. Nous devons leur apporter des assurances, et je sais pouvoir compter sur vous pour accompagner cette démarche. La cohérence, ensuite. L'organisation du déconfinement autour du couple maire-préfet entre en cohérence avec les réalités du terrain. La présentation des cartes d'évolution du virus dans nos départements contribue à cette prise en compte des spécificités locales, loin de toute approche uniforme et peu pertinente. La cohésion j'y faisais référence précédemment. Sachez, mes chers collègues, que, quelles que soient nos sensibilités, nous serons jugés sur notre capacité à entendre le message délivré par les Français, celui de l'unité nationale. Les réflexes politiciens ne feront qu'ajouter de la crise à la crise, soyons-en conscients. La concertation, enfin. C'est le point central du succès du déconfinement : je tiens à vous remercier d'avoir pris en considération les remontées des territoires et associé l'ensemble des élus locaux à ce processus amené à se mettre en place progressivement à partir du 11 mai. Dans la méthode comme dans le fond, monsieur le Premier ministre, je remercie le Gouvernement d'agir avec lucidité et avec humilité. L'expérience de cette crise aura ébranlé nombre de nos préjugés. Le déconfinement est la première étape d'un long chemin qui nécessitera écoute, pédagogie, détermination et courage. Notre groupe sait pouvoir compter sur vous pour mener notre pays sur la voie du redressement sanitaire, économique et social. La parole

et bien qu'en désaccord sur de nombreux points quant à la gestion de cette pandémie par votre gouvernement, j'avais pris la résolution de voter favorablement, comme je l'ai fait d'ailleurs lorsqu'il s'est agi de vous donner les moyens financiers de gérer cette crise. J'avais l'intention de le faire, car je pense que celui qui dirige la manoeuvre par temps difficile doit avoir les moyens d'agir, de s'adapter, bref de bien gouverner. J'avais l'intention de le faire, car vous avez enfin pris la décision de pratiquer une politique intensive de tests que, à mon grand regret, vous n'aviez pas pu ou voulu mettre en place, à l'instar de l'Allemagne, de la Corée ou de Taïwan. J'avais apprécié également votre volonté de remettre à plus tard l'application StopCovid, après la tenue d'un débat. Las ! Les paroles sont une chose, la réalité des actes en est une autre. J'ai été choqué

des parents, vous leur laissez une responsabilité morale importante et ils n'auront pas nécessairement les moyens de faire des arbitrages. Comment feront les maires si 80 % des parents envoient leurs enfants à Cerise sur le gâteau, la carte des départements rouges ou verts relève de la plus grande fantaisie quant aux chiffres qui ont été pris en compte pour définir les différents paramètres.

Pour toutes ces raisons, je me vois dans l'impossibilité de voter favorablement, monsieur le Premier ministre, et je le regrette : il y a trop loin de la parole aux actes. J'espère que le Sénat pourra amender votre texte

car, au-delà de la santé, il pourrait y avoir des conséquences économiques importantes ; j'espère surtout que nos scientifiques nous aideront rapidement à sortir de cette crise majeure.

vous nous présentez, monsieur le Premier ministre, votre stratégie nationale de déconfinement, après l'avoir fait à l'Assemblée nationale devant nos collègues députés le 28 avril dernier. Mais, aujourd'hui encore, il ne s'agit pas d'enrichir votre plan : vous nous demandez de le voter tel quel, comme vous l'avez élaboré. Et même si vous avez organisé, entre-temps, des visioconférences avec les associations d'élus et les partenaires sociaux, vous nous demandez en réalité un vote de confiance. Ce n'est pas notre conception de la démocratie ! La confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Or, monsieur le Premier ministre, vous avez largement entamé votre capital confiance auprès de l'opinion publique. Depuis le début de cette crise, les Françaises et les Français sont assaillis d'injonctions contradictoires sur le port du masque ou encore sur la nécessité de pratiquer ou non des tests. Et l'impression dominante est que vous adaptez votre stratégie non pas à la sécurité sanitaire de chacune et de chacun, mais aux pénuries de matériel de protection ! Il en est de même pour la reprise de l'école, qui paraît plus dictée par la nécessité de reprise économique que par la volonté de faire reculer les inégalités scolaires. Pourquoi, sinon, maintenir les cartes scolaires qui programment des fermetures de classes, un peu partout sur le territoire, dès la rentrée de septembre ? Bien sûr, il existe de nombreuses inconnues concernant le Covid-19 qui ne peuvent vous être reprochées. Chaque jour, nous apprenons de cette épidémie et les chercheuses et chercheurs du monde entier sont sur la brèche. Un traitement sera trouvé, à n'en pas douter, puis un vaccin pour protéger les populations. Ce qui devrait vous faire réfléchir, d'ailleurs, à l'importance vitale du financement de la recherche publique, qui manque cruellement de moyens financiers et humains. Mais, en attendant, il faut faire face et vous avez de lourdes responsabilités dans la gestion de la pandémie, monsieur le Premier ministre. Comme vous l'avez justement souligné, la stratégie de déconfinement passe par le triptyque « protéger, tester et isoler ». Et protéger nécessite notamment le port du masque. Sans revenir sur la gestion des stocks de masques par votre gouvernement et ceux qui l'ont précédé, comment ne pas dénoncer le fait que notre pays soit passé de 1 milliard de masques chirurgicaux et 700 millions de masques FFP2 en 2009 à 145 millions de masques chirurgicaux en 2020 ? L'État n'étant pas en mesure de fournir le nombre de masques nécessaires, ce sont les collectivités qui ont pris le relais. Et aujourd'hui, celles qui ont été les plus réactives sont pénalisées, car elles ne bénéficieront même pas de la prise en charge de 50 % de leur coût par l'État si l'on suit à la lettre vos propos ! Nous demandons que toutes les commandes des collectivités soient prises en charge à égalité, indépendamment de la date de commande. Par ses défaillances, le Gouvernement a mis les collectivités en concurrence. C'est insupportable ! Et, comme l'ensemble des membres de mon groupe, je suis scandalisée de voir que la grande distribution réussit que la puissance publique ne parvient pas à faire. Ainsi, dans ma ville de Gentilly, comme dans beaucoup d'autres sur l'ensemble du territoire, des pharmacies n'étaient toujours pas en mesure, samedi, d'avoir des masques pour les populations Il n'y a aucune raison que les acteurs privés fassent des profits sur la santé et la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes, des personnels médicaux, paramédicaux et ceux du secteur médicosocial Pour nous, les masques doivent être pris en charge comme un matériel médical et remboursé à 100 % par la sécurité sociale au même titre que le sont les tests. Quand le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, ce que nous soutenons totalement, il est de la responsabilité de l'État de garantir le droit au masque gratuit pour toute la population. Et si les masques sont en nombre insuffisant, je ne vois pas comment on peut verbaliser celles et ceux qui n'en portent pas ! Et il y a le même flou concernant la reprise de l'école. Le retour des enfants sur le chemin des écoles est un impératif pédagogique et de justice sociale, mais si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, je partage totalement le refus de l'Association des maires d'Île-de-France de rouvrir le 11 mai prochain les écoles. Quant aux parents d'élèves, ont-ils réellement le choix avec la menace qui pèse sur le chômage partiel le 1 juin ? Mais nous y reviendrons lors de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, tout comme sur la protection juridique des maires. Parler de déconfinement, monsieur le Premier ministre, c'est aussi parler offre de soins, donc capacité d'accueil des patients, nombre de lits et embauches de personnels soignants et non soignants. Vous ne cessez de répéter que l'hôpital a tenu, mais, comme nous l'ont rappelé les docteurs Christophe Prudhomme et Gérald Kierzek, deux éminents urgentistes auditionnés par la commission des affaires sociales, en réalité, il n'a pas tenu ! Il a fallu le confinement général et l'arrêt des activités médicales hors Covid-19 pour passer le pic ! Et pour cause, puisque cette situation de notre système de santé est est le fruit de choix politiques assumés : 4,2 milliards d'euros de moins pour le budget 2020 de la sécurité sociale, dont 1 milliard pour l'hôpital public. Le tout dans un climat de réduction de personnels et de fermetures de lits vingt ans, 100 000 lits ont été fermés, dont 17 500 depuis six ans. Il ne suffit pas de féliciter, dans les discours du Gouvernement, les héros et héroïnes en blouse blanche ; il faut leur donner les moyens humains et financiers d'exercer leur métier. À quand une augmentation de leurs salaires, une revalorisation de leurs métiers, la fin de la précarisation à l'hôpital et dans les Ehpad ? Avec votre gestion calamiteuse du nombre de masques, comment vous faire confiance pour repérer, tester et isoler en dix jours ? Cette crise est terrible : elle est sanitaire, économique, sociale et l'on commence à en ressentir les déflagrations, avec une progression de la pauvreté. Les associations caritatives, les collectivités nous alertent sur l'explosion de l'aide alimentaire. C'est maintenant qu'il faut penser au jour d'après. Il faut plus de justice sociale, revoir totalement la fiscalité pour que chacun contribue à l'effort de solidarité nationale et arrêter d'assécher les caisses de notre système de protection sociale en exonérant de cotisations patronales à tour de bras ! Les aides de l'État doivent être conditionnées à des critères sociaux et environnementaux. Vous ne pouvez continuer à donner des chèques en blanc aux grands groupes, à ceux qui polluent notre planète ! Il faut reprendre la proposition que notre groupe avait avec nos collègues députés communistes : refuser les aides et les prêts aux sociétés qui ont des actifs dans les paradis fiscaux, taxer les dividendes et rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il faut arrêter de détruire le code du travail, de réduire toujours plus les pouvoirs des salariés, en refusant notamment au patronat de déroger à la durée du travail, aux congés payés ou encore au repos dominical Il est temps, monsieur le Premier ministre, de déconfiner la démocratie alors que vous transformez le Parlement en chambre d'enregistrement qui doit vous laisser les pleins pouvoirs pour deux mois supplémentaires. Les parlementaires, pas plus que les élus locaux, ne sauraient être tenus responsables d'une politique décidée sans eux. Crise ou pas, la démocratie exige d'élaborer des solutions avec les élus de la Nation,

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, déconfiner ou ne pas déconfiner, telle est la question Je suis fasciné de découvrir que nous avons autant d'experts pour y répondre sur toutes nos chaînes de télévision : les grands experts, très assurés ; les petits experts, qui manquent d'expérience sur Zoom et dont on ne voit que le nez, le menton et les lunettes en gros plan les soi-disant experts, qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio ; et, enfin, les faux experts qui lancent des craques en espérant faire le buzz. À force de tous les regarder, j'ai découvert un théorème, que je vous propose : plus il y a d'experts, moins on comprend. Heureusement, il reste les politiques ! J'ai suivi le débat à l'Assemblée nationale, mercredi dernier, monsieur le Premier ministre. Il y a là-bas des virtuoses du coronavirus. Ils vous ont expliqué ce qu'il fallait faire hier et ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qu'il faudra faire demain. Je revois encore le professeur Mélenchon, de la faculté de médecine de La Havane, pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d'une voix de stentor : « Il y aura un deuxième pic de l'épidémie, et vous le savez ! » Impressionnant J'étais au bord du Devant tant de recommandations de spécialistes, je n'ose pas vous proposer les miennes, moi qui ne suis qu'un simple médecin épidémiologiste. Je voudrais juste me borner à quelques réflexions sur certaines idées qui me paraissent fausses. La plus absurde, c'est que le libéralisme est la cause de la pandémie. Dans ce pays, où beaucoup préfèrent Robespierre à Tocqueville, où l'on préférera toujours se tromper avec Sartre qu'avoir raison avec Aron, c'est toujours le libéralisme qui porte le chapeau. Même les plus ignares des antimondialistes, des populistes et des complotistes devraient pourtant savoir, puisque même Google le dit, que Périclès, mort de la peste en 429 avant Jésus-Christ, ou Saint Louis, mort du même mal en 1270, n'avaient jamais ne serait-ce qu'entendu les mots de capitalisme ou de libéralisme. Le Covid-19 n'est pas une maladie de la mondialisation ; c'est une maladie tout court. Napoléon disait : « L'Histoire est une suite de mensonges sur lesquels on s'est mis d'accord. » Aujourd'hui, il dirait : « L'Histoire est une suite de mensonges qui ont le plus de . » Il fallait trouver le responsable du complot. Au Moyen Âge, c'étaient la colère divine, les sorcières ou les juifs. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. La vérité est l'exact contraire. La grande nouveauté, c'est que c'est la science qui est aujourd'hui mondialisée. Jamais dans l'histoire on n'a donné une réponse aussi rapide à une nouvelle maladie le génome du virus séquencé en une semaine, les premiers tests produits un mois plus tard, les essais cliniques de traitements et de vaccins déjà par centaines. À ceux qui s'impatientent, il faut rappeler que les épidémies d'avant faisaient cent fois plus de morts, qu'il a fallu des milliers d'années avant que Pasteur, en 1885, ne découvre le vaccin contre la rage et que Yersin n'isole le bacille de la peste, et que c'est grâce à la démocratie libérale et à ses progrès scientifiques qu'elles ont été vaincues comme celle-ci le sera demain. Deuxième idée qui traîne, celle des prophètes, qui nous expliquent que, demain, rien ne sera comme avant. Mais dès qu'on les écoute, on s'aperçoit que leur monde futur est celui qu'ils prêchaient avant : l'avenir radieux avec les lunettes du passé. Ils annoncent des révolutions, mais on s'aperçoit qu'ils profitent de la crise pour recycler des idéologies archidécédées mort du capitalisme, haine de la technique, décroissance, éloge du populisme, retour des frontières, nationalisme. Ils courent les télévisions pour annoncer l'avènement d'un monde nouveau, mais leur besace ne contient que la poussière du prêt-à-penser qu'ils ressassent depuis des décennies. La réalité, c'est que personne n'a jamais vu demain. C'est à nous de préparer l'avenir, et il sera sans doute différent. Mais, ce qui est certain, c'est qu'il ne ressemblera sûrement pas à un des thèses de Karl Marx, de Maurras ou de Malthus. Troisième ineptie : les régimes autoritaires seraient les grands gagnants de cette pandémie, car les plus efficaces. C'est le contraire qui est vrai. La cause de la maladie est le virus. La cause du drame est le régime chinois, qui a caché la vérité pendant un mois. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui 25 000 morts en France et des centaines de milliers dans le monde. Les seuls pays qui s'en sont bien sortis sont les quatre démocraties asiatiques : Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud, qui bénéficiaient d'expériences antérieures. J'espère que personne ne va me dire : « Et la Chine ? La Chine qui annonce 4 500 morts sans avoir jamais expliqué à quoi servaient les 50 000 urnes funéraires livrées en urgence, de nuit, dans la seule ville de Wuhan. La Chine dont on ne connaîtra le nombre de morts qu'un jour lointain, comme on n'a connu les 40 millions de morts du Grand Bond en avant que trente ans plus tard, à la mort de Mao. Quant aux populistes en Occident ? Trump, qui restera comme le président du, Bolsonaro, qui laisse s'infecter sans protection les habitants de ses bidonvilles, et Johnson, sauvé de peu de ses propres théories sur l'immunité et dont le pays détient désormais la palme européenne des victimes. Je préfère l'exemple de l'Allemagne démocratique. C'est bien sûr un peu irritant, ces Allemands qui savent toujours où sont rangées les affaires. Mais attention : d'abord, l'Allemagne nous suit de dix jours dans l'épidémie et ses chiffres montent ; ensuite, les résultats allemands sont, hélas, beaucoup plus proches de ceux du reste de l'Europe que de ceux C'est bien dans les démocraties d'Asie du Sud qu'il nous faudra chercher les exemples si nous voulons réussir le déconfinement, et non pas chez les dictateurs. Vous vous apprêtez, monsieur le Premier ministre, à prendre la plus grande décision de cette crise, parce que le déconfinement sera beaucoup plus difficile que le confinement. Vous serez tenté de le faire très prudemment. D'abord parce que, dans nos régimes libéraux, qui s'attachent à rendre impossibles leurs propres décisions, les épées de Damoclès politiques, juridiques et médiatiques vous menaceront à la moindre erreur- les sycophantes ont déjà ouvert leurs dossiers. Mais votre Rubicon est là et vous n'avez d'autre choix que de le franchir sans trembler. Jusqu'à ce jour, entre laisser mourir des hommes et suspendre l'économie, nous n'avons pas hésité et nous avons choisi le confinement. Le 11 mai, en ouvrant les rues, les maisons, les entreprises et les administrations, ne laissons personne dire que nous ferions le choix inverse, celui de l'économie contre les hommes. Au contraire, poursuivre le confinement ou déconfiner trop timidement ferait aujourd'hui beaucoup plus de victimes. D'abord, les victimes, bien plus nombreuses qu'on ne le croit, d'autres pathologies, qui, depuis deux mois, ne se soignent plus. Ensuite, parce qu'une crise économique- et celle qui vient sera l'une des pires -fait bien plus de victimes que le virus, même si le fait de ne pas pouvoir les chiffrer permettra à tous ceux qui n'ont rien compris à l'économie et qui ne l'aiment pas- ils sont nombreux en France -de vous accuser de préférer les profits à la santé de nos concitoyens. Il faut ouvrir les portes et le faire sans hésiter. Et cela veut dire faire confiance aux Français. Ils ont montré- personne ne l'aurait parié -qu'ils étaient capables, aussi bien que des Coréens ou des Allemands, de respecter un confinement drastique. Ils ont compris les gestes, la prudence et la distanciation. Ils ont aussi compris les risques, et c'est d'ailleurs pour cela que, s'ils souhaitent le déconfinement, ils le redoutent en même temps. Il y aura des bosses sur la route, monsieur le Premier ministre, mais il faut prendre la route. Richelieu disait : « Il ne faut pas tout craindre, mais il faut tout préparer. » C'est la tâche qui vous attend aujourd'hui, c'est la tâche qui nous attend tous.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, je voudrais commencer mon propos en remerciant l'ensemble de celles et ceux qui font vivre notre pays au quotidien,

vous êtes aux avant-postes et vous faites le. Bien entendu, cette sympathie et cette compréhension n'emportent pas systématiquement adhésion à toute l'action qui est menée et c'est le rôle du Parlement, justement, que de se montrer critique, de contrôler l'action du Gouvernement et d'examiner les textes qui lui sont soumis. Au demeurant, il travaille lui aussi dans des conditions extrêmement difficiles et contraintes. Pour autant,

S'agissant des tests, la problématique est la même. Cette semaine, les annonces faites par les grandes chaînes de distribution n'ont rien arrangé à l'affaire.

Cette communication est désastreuse pour beaucoup d'entre eux. Davantage- et vous leur avez en partie répondu -s'inquiètent en disant : « On fait confiance aux commerçants pour rouvrir, mais on ne fait pas confiance aux officiants des cultes pour ouvrir de petites églises, de petits temples, de petites mosquées ou de petites synagogues, ici ou là dans nos provinces.

prééminente et tenir compte de ce qui s'est passé, car les Français n'accepteront plus, dans leur grande majorité, qu'on donne beaucoup d'argent aux grandes entreprises sans qu'ils puissent bénéficier d'un retour. S'agissant de la gouvernance mondiale, puisque vous avez évoqué ce point au début de votre propos, cette pandémie est mondiale et l'on a vu la faillite des grandes institutions de l'après-guerre : l'ONU, l'Europe, le G7, le G20. Nous n'avons pas été en mesure d'apporter des réponses collectives. À l'évidence, il faudra repenser rapidement notre participation aux instances mondiales.

d'abord, c'est celle que nous devons aux Français ; c'est l'exigence démocratique. En ces temps de crise, la démocratie n'est pas une gêne ou un obstacle : c'est une ressource.

Notre bienveillance, donc, vous l'avez. Mais la confiance que vous nous demandez cet après-midi, nous ne pouvons pas vous l'accorder aussi facilement, pour plusieurs raisons. La première est que nous ne pouvons plus vous croire sur parole, parce que cette parole a donné lieu à trop de contradictions, à trop de contre-vérités, parfois, aussi, sur ce qui constitue d'ailleurs

Vous auriez dû dire dès le départ qu'il y avait un problème de pénurie. Les Français ne sont pas des sots : ils s'en sont rendu compte. Et c'est ce qui a écorné la confiance que vous estimiez, il y a quelques instants, absolument nécessaire en vue du déconfinement.

des ratés, des lenteurs, des lourdeurs. À l'Assemblée nationale, vous avez plaidé l'humilité ; ... Eh oui ! ... c'est un mot que vous n'avez pas prononcé aujourd'hui

Oui, il faut déconfiner. Oui, nous sommes favorables au déconfinement, parce que les inconvénients du confinement sont désormais, y compris en termes sanitaires, supérieurs à ses bénéfices. Mais ce plan de déconfinement ne saurait être un pari à quitte ou double Je vous ai entendu, à l'Assemblée nationale, prononcer une phrase clé qui résume peut-être votre climat intérieur, en tout cas la tonalité de l'ensemble de votre discours- je vous cite, mot à mot : « Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas.

qu'il s'agit sans doute, de toutes les décisions que vous avez prises, de la plus difficile et de la plus grave. Je ne dis pas qu'elle est simple ; je dis seulement que nous aurions pu, à l'instar d'autres pays,

trouver. Vous pouvez compter sur notre bienveillance. Mais nous avons des doutes. C'est la raison pour laquelle nous allons très majoritairement, massivement même, nous abstenir. Vous pouvez compter sur nous pour améliorer le texte

concourir à l'application des décisions de l'État. En tout cas, comme je l'ai dit, nous restons disponibles pour améliorer ce texte. Sans méconnaître la difficulté de votre situation- vous n'avez pas choisi la date du 11 mai -, je pense qu'il faut impérativement, désormais, faire en sorte que la France puisse retrouver le peloton de tête des pays qui, dans le monde entier, ont su combattre efficacement cette pandémie, en essayant de casser les chaînes de contamination, ce que jusqu'à présent nous n'avons pas fait. Nous avons freiné l'épidémie, mais nous ne lui avons pas cassé les reins. La

perdant leur vie pour certains- je veux leur rendre hommage -, ainsi qu'aux millions de Français qui sont chez eux, confinés. Le pays tout entier est mobilisé pour faire face, et chacun doit assumer sa responsabilité.

et de travailler, mais qui ne doit pas provoquer un effondrement économique. La grande faucheuse sanitaire ne doit pas se muer en une grande faucheuse sociale.

La seule certitude que nous avons aujourd'hui est que nous allons devoir vivre de longs mois avec ce virus. Ce constat étant fait, le défi du déconfinement est une étape cruciale. Nous savons qu'un déconfinement raté serait le prélude à un reconfinement assuré. Une deuxième vague réduirait à néant les efforts fournis jusqu'à présent et viendrait heurter de plein fouet un système de santé déjà très affaibli par la première vague. Le déconfinement est un pari à haut risque, monsieur le Premier ministre. La date du 11 mai a été fixée, mais cette annonce avait-elle été vraiment préparée par un travail de fond de votre gouvernement, dans une logique de rétroplanning ? Permettez-moi, sur ce

au besoin de clarté de la population doit être la première préoccupation de votre gouvernement : il faut en finir avec les injonctions contradictoires que nous connaissons depuis plusieurs mois. J'ai en mémoire vos propos rassurants, le 27 février, quand vous aviez réuni à Matignon les présidents de groupes et les patrons de partis. Nous étions sortis de cette réunion, sinon rassurés, en tout cas rassérénés. Les injonctions contradictoires, les ordres et les contre-ordres ajoutent de l'anxiété à une période qui n'en manque pas. Mais, par-dessus tout, cela fait courir un risque sanitaire. Il faut que les règles édictées soient comprises et partagées, afin d'éviter une deuxième vague. une illustration, cela a déjà été dit : le manque de garanties concernant l'accessibilité des masques aux Français, et l'absence de prise de position du Gouvernement sur la gratuité. Avec le temps qui passe, les Français se sont rendu compte que, contrairement à ce qui était avancé, les masques ne sont pas inutiles s'ils deviennent une protection collective et massive. Nous avons donc du mal à comprendre pourquoi les masques seraient obligatoires à l'école et dans les transports alors qu'il n'existe aucune obligation de les porter au travail ou dans les lieux publics. Nous souhaitons avoir des éclaircissements sur ce point.

actuel, n'a pas de sens. L'État doit prendre ses responsabilités et ne pas craindre de poursuivre ses réquisitions pour permettre à l'ensemble des Français d'être correctement protégés dès qu'ils entrent dans l'espace public. Quant aux tests, nous demandons des points d'étape réguliers sur leur nombre et les garanties entourant leur disponibilité. Je ne vous rappellerai pas, monsieur le Premier ministre, qu'il y a encore à peine un mois nous étions à 5 000 tests par jour 5 000 tests par jour ! Vous nous annoncez 100 000 tests par jour le 11 mai ? Tant mieux ! Mais nous serons là pour vérifier que cet engagement sera bien respecté. bien respecté. La prise en charge de l'isolement des personnes malades doit également être assumée par l'État lorsque celles-ci ne disposent pas d'un lieu où s'isoler. La question de la restriction des libertés publiques proportionnée à l'urgence doit elle aussi être traitée avec le plus de clairvoyance possible. S'il faut donner les moyens aux brigades sanitaires de faire leur travail, il convient de repousser les dispositifs inefficaces et dangereux pour la liberté des Français, comme l'application StopCovid. La ligne de crête est étroite, mais la République doit veiller à ne pas céder à la panique et continuer à garantir les libertés fondamentales. Vous sembliez douter, à l'Assemblée nationale, de la pertinence de ce dispositif.

Si ce conseil est consultatif, il ne doit pas devenir décoratif. Pour ne pas avoir suivi ses recommandations concernant les écoles, vous finissez par créer un doute dans l'esprit des Français. L'école ne doit pas devenir le symbole de l'échec du déconfinement. Or la reprise progressive de l'école sur une base volontaire traduit l'incertitude relative aux conditions de sécurité sanitaire. Le risque que fait courir une reprise anticipée aux enseignants et aux élèves est trop grand ; il est urgent d'attendre pour que l'école ne devienne pas le creuset d'une nouvelle catastrophe sanitaire. De nombreux maires s'inquiètent de la faisabilité de cette reprise. Plusieurs centaines d'entre eux vous ont écrit et ont demandé au Président de la République, hier, de repousser la réouverture des écoles. Quelle réponse leur apporterez-vous ? L'État ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en faisant peser la décision de la rescolarisation sur les parents et la décision de la réouverture sur les maires seuls. L'école à la carte, à pile ou face ou sur un coup de dé n'est pas conforme au principe républicain d'égalité. Vous n'avez pas anticipé le désarroi des parents, des enseignants, des élus. Dans ce contexte très particulier, il conviendra de clarifier les conditions dans lesquelles la responsabilité des maires

Prolongeons le chômage partiel ; arrêtons de précariser les chômeurs et abrogeons définitivement votre réforme injuste de l'assurance chômage ; engageons des négociations salariales ; créons le revenu de base ; abandonnons votre projet mortifère de réforme des retraites retraites ! Ces mesures prioritaires avaient selon nous leur place dans le projet de loi examiné ce soir. Ce texte aurait dû être un projet de loi d'urgence sanitaire et sociale. Malheureusement, il n'en est rien. Vous le voyez, nos craintes sont nombreuses. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de développer bien d'autres sujets que nous évoquerons à l'occasion de questions complémentaires. En particulier, l'équilibre fragile entre la sécurité sanitaire des Français et la protection de leurs libertés individuelles sera au coeur de notre débat. Monsieur le Premier ministre, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour accompagner les Français. Nous avons d'ailleurs adopté les deux projets de loi de finances rectificative. Mais l'exercice, aujourd'hui, est différent, face à la crise. Aujourd'hui, vous nous demandez de vous accorder notre soutien. le soutien se construit dans la confiance : confiance dans la gestion passée, confiance dans les choix à venir, confiance dans les moyens développés et déployés.

monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, au nom du groupe du RDSE, je voudrais tout d'abord avoir une pensée compatissante pour tous nos compatriotes emportés par le Covid-19, pour leurs familles, pour leurs amis, pour leurs proches, qui, bien souvent, n'ont pu se recueillir comme ils l'auraient souhaité. À l'évidence, nous avons plus que jamais besoin d'humanité, alors que nos sociétés modernes sont devenues des monstres de complexité et de technologie, innervés de connexions innombrables et mondiales. Pour autant, le progrès technique n'empêchera jamais le drame intime dans toute sa crudité, car nous demeurons ontologiquement fragiles. Trop sûrs de notre maîtrise de la nature, nous en oublions notre finitude. Le rappel actuel est violent, mais c'est aussi dans la science que nous plaçons aujourd'hui nos espoirs, saluant à juste titre- mon groupe s'est une nouvelle fois -le travail exceptionnel de l'ensemble du personnel médical et des chercheurs. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit la semaine dernière et rappelé il y a quelques instants : face à la situation exceptionnelle que connaît notre pays, le confinement reste le meilleur outil pour contenir l'épidémie, au prix d'efforts intenses de chacun, d'un sens civique aigu, mais aussi de conséquences vertigineuses- la crise économique et sociale frappe déjà. Oui, les contaminations reculent, les admissions en réanimation diminuent. Néanmoins, le combat sera encore long. Aucun relâchement n'est possible si nous voulons éviter une seconde vague. Comme le dit notre collègue le docteur Véronique Guillotin, nous devons apprendre à apprivoiser ce virus que seul le vaccin pourra tuer. Pour autant, le prix du confinement est élevé pour nos compatriotes : isolement social, pertes de revenus, faillites d'entreprises, aggravation des fractures sociales et territoriales, la liste est longue, car notre pays, comme les autres, s'est quasiment arrêté du jour au lendemain. Déconfiner est donc une nécessité absolue, pour relancer notre économie, bien sûr, donner les moyens aux services publics de fonctionner et, surtout, répondre aux angoisses de notre inconscient collectif. Plus que jamais, la solidarité doit être au coeur de notre action collective. action collective. Le déconfinement suppose donc humilité et responsabilité. De ce point de vue, monsieur le Premier ministre, mon groupe partage votre approche à la fois pragmatique, progressive et territorialisée. Les détails peuvent, eux, toujours être débattus, mais la préservation de nos libertés ne se discute pas. Nous sommes sur un fil- c'est votre expression -dans la perspective du 11 mai. Les conditions sont drastiques- vous les avez rappelées : capacité à tester massivement, moindre circulation du virus, état des hôpitaux, baisse du taux de contamination par malade, le fameux R0. Nous mesurons pleinement la difficulté et la gravité des décisions à prendre en vue de préserver la continuité de notre pacte républicain. À ce titre, je voudrais insister sur un point : aucune instance, si éminente soit-elle, ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité politique légalement formée. Les avis du conseil scientifique sont certes indispensables, mais ils ne sont pas contraignants. Leur publication en temps réel doit absolument être mise en perspective avec le temps de la décision politique. Monsieur le Premier ministre, si nous souscrivons à votre objectif et à votre approche, de nombreuses incertitudes persistent. J'ai d'ailleurs une modeste suggestion à vous faire quant à la carte publiée chaque jour n'oubliez pas d'y inclure tous les territoires ultramarins de la République, comme Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et pas seulement les départements d'outre-mer ; je sais que nos concitoyens des collectivités d'outre-mer y seront sensibles. Plus largement, les élus locaux, les maires en première ligne, ont admirablement rempli leur rôle, y compris ceux qui vont passer la main d'ici peu. De nombreuses initiatives locales ont permis de conserver un lien social de qualité au plus près de nos concitoyens, et en particulier des plus fragiles, malgré la complexité normative. Tous attendent maintenant que soit fixée la suite du calendrier électoral, sans oublier qu'il faudra aussi rapidement stabiliser les exécutifs intercommunaux pour solidifier leur action. Je voudrais également saluer toutes les collectivités qui se sont engagées pour soutenir financièrement les PME en difficulté, en dépit d'un cadre juridique inextricable, sur lequel nos collègues Raymond Vall et Josiane Costes ont donné À l'approche du 11 mai, la réouverture des écoles est une autre source d'inquiétude, pour les élus comme pour les enseignants, parents et enfants. La diffusion des protocoles sanitaires ne devrait ne devrait y remédier qu'en partie, car, vous le savez, la question des responsabilités administrative et pénale des élus cristallise l'attention. Nous aurons tout à l'heure ce débat, lors de la discussion du projet de loi. Mais je tiens d'ores à dire qu'il n'est pas question pour mon groupe de laisser les élus locaux supporter seuls le poids de responsabilités qui ne sont pas les leurs. Quelques mots encore sur un sujet que vous avez brièvement évoqué, celui de la culture, cher notamment à Françoise Laborde. Ce secteur, qui contribue tant à notre rayonnement et à notre vie sociale, est évidemment très inquiet, sachant que le risque de déstabilisation durable est réel. Les professionnels attendent de la visibilité, mais espèrent aussi un protocole sanitaire précis pour préparer la reprise de leurs activités. Monsieur le Premier ministre, il est toujours plus facile d'être dans la posture du commentateur que dans celle du décideur. Il sera toujours temps, dans les prochains mois, d'analyser les dysfonctionnements de l'action publique ; mais, si nous le faisons, c'est toujours, pour

La discussion du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire permettra d'aborder en profondeur de nombreuses questions qui interpellent nos compatriotes. Mon groupe, par la voix de Maryse Carrère, rappellera son attachement viscéral aux libertés publiques, que même une grave épidémie ne saurait mettre en suspens. Pour l'heure, après vous avoir attentivement écouté et vu les enjeux pour notre pays et nos concitoyens, une large majorité du groupe du RDSE approuvera votre déclaration. La parole est

à l'occasion de cette réponse, l'ensemble des sujets que vous avez évoqués. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des orateurs pour leurs propos. Permettez-moi de saluer, au premier rang d'entre eux, ceux qui ont relevé la difficulté du moment et exprimé leur soutien au Gouvernement. Sans répondre sur tous les sujets, je voudrais, avec le président Requier, faire le constat que la critique est facile et l'art difficile- c'était le sens de votre propos, monsieur le sénateur. Je ne dénigre pas ceux qui critiquent ; il se trouve qu'il est souvent plus facile d'avoir un avis sur une décision que quelqu'un d'autre prend.

de prendre des décisions et de les présenter. Pour illustrer néanmoins la difficulté de cette tâche, je voudrais utiliser la question qui a été posée par le président Kanner à propos de l'application StopCovid.

densité et d'anonymat. Vous êtes dans une rame de métro, avec quarante personnes ; vous ne les connaissez pas, elles ne vous connaissent pas, elles peuvent être près de vous, même si la distanciation physique s'impose en toutes circonstances.

et vous pourriez informer de façon anonyme, sans savoir qui était en face de vous, quelqu'un qui serait resté à moins d'un mètre de vous pendant trois minutes, et ce grâce à cette connexion Bluetooth sur laquelle les scientifiques et les techniciens travaillent. Vous le voyez, dans ce cas-là, et sans doute dans ce cas-là seulement, cet

car techniquement, elle n'avait pas obtenu toutes les validations requises, et que nous n'allions pas nous poser la question de savoir s'il fallait l'utiliser dès lors qu'elle n'était pas prête, car les questions théoriques, c'est bien, mais pour l'instant, je préfère me poser des questions pratiques

nous ne sommes plus en mesure, dans un tel département, de garantir la remontée de l'ensemble des chaînes de contamination. Ce jour-là, on a un vrai problème dans le département ! Je suis obligé d'y penser.

progressivement mis en place sont de plus en plus protecteurs. On trouve toujours derrière la réglementation sanitaire des considérations qui ont été jugées par les pouvoirs en place excellentes, et je ne les conteste pas. J'observe que J'observe que vouloir lever, et rapidement, les dispositifs un par un est un exercice qui, lui aussi, renvoie à une certaine forme d'humilité- croyez-moi

donner quelques directions vagues, ou claires, mais formulées en termes de principes, c'est à coup sûr, vous le savez, s'exposer à la critique de ceux qui diront : « Vous avez formulé quelques principes clairs, mais sur le terrain, vous laissez les gens se débrouiller.

va être très difficile, mais dans beaucoup d'autres, tout va bien se passer- j'en ai la conviction. J'observe d'ailleurs avec intérêt qu'un certain nombre de ceux qui critiquent ces éléments

Je ne veux pas me comparer à des chefs d'État qui dirigent de grandes puissances outre-Atlantique- je n'en ai ni le physique ni le caractère -, mais

maintenant procéder au débat interactif sous la forme d'une série de quinze questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

à M. Xavier Iacovelli. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays, les maires et les élus locaux sont en première ligne pour protéger nos concitoyens et mettre en oeuvre les mesures d'urgence permettant de faire face à cette situation inédite. En tout état de cause, celle-ci laissera des traces, tant elle a bouleversé notre quotidien, frappé celles et ceux qui nous entourent, fortement touché nos commerçants, artisans, indépendants et les familles les plus précaires. Dans ce contexte, les maires sont au plus près des réalités du terrain et en contact permanent avec nos concitoyens pour répondre à leurs attentes et à leurs inquiétudes. Ils sont, et je reprends vos mots, monsieur le président, « à portée d'engueulade » de leurs administrés. Ces mêmes élus locaux auront pour mission d'assurer la réouverture des écoles à compter du 11 mai prochain, telle qu'elle a été prévue par le Gouvernement. Dans ce cadre, et vous l'avez rappelé, monsieur le Premier ministre, la protection de nos enfants est la priorité. Les conditions de sécurité sanitaire doivent être scrupuleusement respectées, et nous pouvons compter sur le dévouement et le travail acharné des maires pour les mettre en oeuvre. Cette priorité, selon nous, va de pair avec le renforcement de la protection juridique des maires et des élus locaux dans le cadre des opérations de déconfinement et, en particulier, dans le cadre de la réouverture des écoles. Oui, vous l'avez rappelé, monsieur le Premier ministre, la loi Fauchon protège déjà les élus. Mais ils ont aussi besoin d'être rassurés par l'État. Il y va de la confiance et de la réussite de ce déconfinement. C'est pourquoi la majorité du groupe La République En Marche a déposé un amendement allant dans ce sens et se félicite de l'adoption d'un amendement similaire du rapporteur. Étant toutes et tous en lien avec les élus de nos départements, nous entendons leurs inquiétudes légitimes et sommes particulièrement déterminés à y apporter une réponse concrète. Ma question est donc la suivante, monsieur le Premier ministre : quelles seront les réponses du Gouvernement face aux attentes des maires et des élus locaux, partenaires essentiels de l'État dans la crise que nous traversons ? je vous remercie les maires doivent pouvoir prendre pour leur commune les décisions qui sont nécessaires au déconfinement, sans crainte de voir leur responsabilité pénale engagée. Ainsi que je l'ai rappelé la semaine dernière à M. le sénateur Bockel, les règles du code pénal qui sont prévues pour retenir la responsabilité pénale en cas d'infraction involontaire sont très très restrictives. Elles reposent sur la recherche d'un comportement sciemment dangereux, d'une prise délibérée de risque, au mépris de la sécurité d'autrui. Ces dispositions font en outre l'objet d'une approche très encadrée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui retient la nécessité de la nécessité de prendre en compte les compétences propres à chacun des élus concernés, d'une part, et l'état des connaissances générales sur tel ou tel domaine, d'autre part, le tout pour apprécier l'existence d'une éventuelle faute. Ce cadre juridique étant général, je ne vois pas comment un décideur, un élu qui donnerait des instructions afin d'assurer notamment le respect des dispositifs barrières pourrait voir sa responsabilité engagée. Il nous appartiendra toutefois de vérifier si la codification de la jurisprudence est nécessaire. Il s'agirait, en opérant ainsi une clarification et une réaffirmation du droit, de prévenir une incertitude qui pourrait être préjudiciable à la prise des décisions qu'imposent les circonstances. Dans ce cadre-là, nous sommes évidemment tout à fait décidés à conduire ce travail avec le Parlement.

la crise que nous traversons est sans précédent. Elle est sanitaire, mais aussi économique et sociale, et même simplement alimentaire. La pandémie et le confinement ont rendu plus visibles que jamais les inégalités rongeant notre société. Pour les plus fragiles, l'épreuve traversée a été plus redoutable encore enfants privés d'un repas à faible coût à la cantine, foyers confrontés à une quasi-famine, étudiants, migrants, mineurs non accompagnés, chômeurs, sans-abri, travailleurs précaires, familles monoparentales, pour qui il s'agit moins de vivre que de survivre Le déconfinement en soi n'effacera pas magiquement ces inégalités criantes ni ne corrigera leurs effets aggravés par cette crise. Il ne s'agit pas seulement de panser les blessures immédiates, de répondre à l'urgence, mais il convient, pour une fois, d'appréhender la question sociale et celle des inégalités dans leur globalité et sur le long terme. Le déconfinement doit être accompagné d'un plan d'urgence sociale redonnant à l'État-providence tout son rôle. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures sociales concrètes et immédiates d'envergure comptez-vous mettre en oeuvre ?

je veux saluer ici l'action. Ils sont aux avant-postes, au contact direct de la population, et, comme l'a dit le Premier ministre, avec les préfets, c'est sur eux que repose le succès du déconfinement. C'est grâce à eux que les déchets sont collectés, que l'eau est distribuée, que les repas sont servis aux plus fragiles. C'est aussi grâce à eux que, demain, les enfants retourneront à l'école avec le plus de sécurité possible. Le Gouvernement a raison de leur faire confiance pour organiser la réouverture des classes, qui est si indispensable à la reprise de notre pays comme à nos enfants.

pouvez-vous rassurer les maires sur la date prévisible d'installation des conseils municipaux qui ont été élus au premier tour ?

de conseillers communautaires qui n'ont pas été définitivement élus au premier tour et dont la légitimité, bien que n'étant pas contestable, puisque la loi a prévu la prorogation de leur mandat, les place dans une situation différente,

Animé par notre collègue Jacques Grosperrin, ce groupe, dont je salue l'excellent travail, a émis onze préconisations, lesquelles ont été rendues publiques, sur le fondement de deux prérequis : l'avis de la communauté scientifique sur la situation sanitaire et ses recommandations, l'urgence d'une concertation avec les acteurs de terrain, notamment les collectivités territoriales. Interpellé par le refus de plusieurs maires, et pas uniquement dans les départements rouges, écouté les familles et des enseignants, le groupe Union Centriste veut des réponses précises, d'abord sur les risques épidémiologiques, les services pédiatriques dans toute la France se faisant l'écho d'un nombre anormalement élevé de pathologies cardiaques affectant des enfants, lesquelles pourraient être liées au Covid-19. Avez-vous des études sur ce sujet, mais aussi sur la contagiosité des enfants ?

et juridique est en effet posée. Sur l'initiative d'Hervé Maurey, notre groupe a d'ailleurs le premier soulevé ce sujet. J'ajoute que certains maires se sentent fragilisés par une élection municipale non achevée.

des enfants en situation de handicap ? Le flottement du début a laissé place à un peu plus de méthode, mais nous avons tous le sentiment d'avancer à marche forcée, avec le 11 mai en ligne de mire.

Vous avez annoncé un certain nombre de décisions, mais pas toutes les décisions. Il reste de mon point de vue trop de flou pour que le compte à rebours qui va nous conduire dans quelques jours au 11 mai soit suffisant

De mon point de vue, dans les départements verts, le travail effectué entre les mairies et l'éducation nationale doit permettre de rouvrir partout les

gravirons la deuxième marche, lorsque, je l'espère, nous aurons relancé notre économie, rouvert notre pays, et que nous aurons montré notre capacité à maîtriser l'épidémie, la distinction entre vert et rouge pourra donner lieu à d'autres différenciations. Au fond, cet indicateur, qui nous permet de savoir si les choses sont parfaitement sous contrôle ou si la menace reste très présente, nous permettra de différencier au fil du temps les mesures qui peuvent être prises dans les départements verts et celles qui ne peuvent pas l'être dans les départements rouges. Vous avez ensuite évoqué le système d'information. Notre objectif est évidemment qu'il soit prêt.

les aider, par exemple, à mieux réguler les arrivées dans les transports ou les horaires de travail ? Nous essaierons de le faire, dans la limite des instruments juridiques à notre disposition. Il n'est en revanche pas prévu à ce stade- je n'en ai parlé ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat -une quelconque attestation pour avoir accès aux transports publics.

des annonces de Mme Pénicaud sur la dégressivité du chômage partiel à partir du 2 juin. La ministre a annoncé que, à partir du 2 juin, le dispositif de chômage partiel serait moins « généreux ». Je ne sais pas si j'aurais employé ce mot si j'avais été à sa place et je ne sais pas si les Français ont eu l'impression de bénéficier d'une générosité quelconque quand ils ont été mis au chômage partiel, mais bref ... Cette remarque est incidente. La ministre a également dit que les parents devront fournir une attestation lorsqu'ils seront contraints de continuer à garder leurs enfants.

Ces derniers jours, un débat s'est engagé au sein de la société et de notre assemblée sur la ligne de crête qui existe entre la protection des libertés individuelles et la protection de la santé publique. L'efficacité du traçage des cas contacts dépendra en effet de multiples facteurs, dont l'adhésion de la population et des professionnels de santé de première ligne. Or des questions restent encore aujourd'hui en suspens concernant le respect de la vie privée, la protection des données individuelles et du secret médical pour les médecins. Pour ma part, je m'interroge sur la cohérence du discours des pouvoirs publics : d'un côté, la restriction de certaines libertés publiques est présentée comme indispensable pour lutter contre le Covid-19, de l'autre, l'extension du port obligatoire du masque, justifiée médicalement, est laissée dans le flou. D'autres pays ont diffusé des messages clairs à ce sujet. Je pense par exemple au Luxembourg, où le masque est depuis aujourd'hui obligatoire dans toutes les situations- transports en commun, magasins -, partout où une distance de 2 mètres ne pourra être respectée. En France, ce message me semble brouillé. Le masque est recommandé, mais pas obligatoire, sauf dans les transports publics et dans les commerces qui le demandent. Or on sait qu'une information précise conditionnerait le respect des consignes et apaiserait les tensions dans l'espace public. On sait aussi que l'efficacité

en un seul semestre, notre pays aura connu trois périodes totalement distinctes, et ô combien singulières : celle d'avant le confinement, où on ignorait à peu près tout du Covid-19 ; celle du confinement, à partir du 17 mars, où, à juste titre, l'impératif sanitaire l'a emporté sur toute autre considération ; puis, à partir du 11 mai, la période que nous appelons, un peu vite sans doute, celle du déconfinement, période inédite durant laquelle notre pays devra conjuguer cette fois l'impératif sanitaire et l'impératif économique et social. Il faut le dire avec gravité, nous abordons des terres inconnues. Les amortisseurs et les dispositifs d'aide publique ont permis d'éviter l'effondrement de notre appareil productif. À présent, il faut impérativement favoriser la meilleure transition pour qu'une majorité de salariés passe du chômage partiel au travail, sans passer par la case Pôle emploi. C'est un enjeu considérable, qui exige la confiance de tous, celle des Françaises et des Français, celle des entrepreneurs et celle des partenaires sociaux.

quelle méthode de dialogue social envisagez-vous avec les partenaires sociaux ? Les sujets à aborder sont nombreux : l'Unédic, les secteurs à l'arrêt- je pense au tourisme, à la culture, aux intermittents du spectacle, aux cafés et aux restaurants

Vous savez aussi, vous en avez entendu parler, que la maladie de Kawasaki touche actuellement pas mal d'enfants sur le territoire national. La semaine dernière, 23 enfants atteints de cette maladie avaient été hospitalisés

des solidarités et de la santé. Merci, monsieur le président Alain Milon, pour votre question. Vous l'avez dit vous-même, Mary Mallon, cette Américaine, était porteuse de la maladie et l'a transmise sans le savoir et sans le vouloir.

Pourtant, je sais que si je vous disais que la culture n'est pas un supplément d'âme, mais qu'elle est notre âme, vous seriez d'accord. Si je vous disais que la culture dans sa diversité est ce qui nous permet de rêver, d'imaginer, de connaître, de nous rencontrer, de nous projeter, de chercher du sens et d'en donner, vous seriez d'accord aussi. Si je vous disais que tout cela s'est particulièrement démontré pendant cette crise, où les artistes, professionnels et amateurs, celles et ceux qui nous informent, nous apprennent ou nous divertissent ont été indispensables à notre vie confinée pour tenir ensemble et individuellement, vous seriez encore d'accord.

au-delà des mois où toute activité aura été impossible. Je vous demande également des mesures d'urgence pour tous les travailleurs en contrat court, qui ne se verront proposer aucun des emplois que les secteurs d'activités culturels offrent en temps normal, afin de maintenir leurs droits d'indemnisation et leurs moyens d'existence.

vous avez raison, les acteurs de la culture, notamment les artistes, jouent un rôle considérable dans notre pays et pour nos compatriotes. Ils ont joué un rôle considérable pendant le confinement et ils vont jouer un rôle considérable pour la sortie de crise.

toute l'économie bénéficient aussi au secteur culturel : les prêts garantis par l'État, l'accès au chômage partiel, le report des charges sociales et fiscales,

du ministère de l'économie et des finances et sous l'autorité du Premier ministre, bâtissons des solutions d'avenir pour nous assurer que cet écosystème si important puisse être sauvé et que nous puissions continuer de nous appuyer

Monsieur le ministre, je vous ai posé une question précise. Je sais que vous êtes suspendu à la parole du Président de la République, mais nous sommes au Parlement, et je ne doute pas que vous savez aujourd'hui si vous allez accorder cette année blanche

mois de mars, la commission des affaires économiques attirait déjà l'attention du ministre de l'économie sur un point qui est vite apparu comme essentiel pour réussir la reprise économique, à savoir la responsabilité des chefs d'entreprise. Au regard du peu de certitudes que nous avons sur le Covid-19 et sa propagation, force est de constater que le risque de contamination sur le lieu de travail pourrait encore exister malgré le respect des consignes sanitaires. Les chefs d'entreprise et les salariés devront « vivre avec », selon votre expression, monsieur le Premier ministre. Nous appelons bien sûr à la reprise de l'activité économique, et nous affirmons ici que la protection des salariés est prioritaire, mais la confiance des employeurs pourrait aussi être entamée si, en dépit des efforts fournis, de la bonne application des consignes et de la concertation avec les partenaires sociaux, leur responsabilité pouvait encore être engagée. Je vous ai bien entendus, madame la garde des sceaux, monsieur le Premier ministre, mais, avec la loi Fauchon, il existera toujours une possibilité qu'un juge considère que toutes les mesures nécessaires n'ont pas été mises en oeuvre, puisque cette loi précise que ces personnes seront pénalement responsables si elles ont commis une faute caractérisée. Il faut donc bien que le juge caractérise cette faute ; or vous savez que, en la matière, la jurisprudence a fait des allers et retours. À la demande des syndicats, le ministère du travail a publié hier un manuel général de déconfinement. Ce manuel est bienvenu, mais il n'est qu'indicatif, car, à moins que vous nous disiez le contraire, il n'a pas de caractère juridique avéré de nature à protéger les chefs d'entreprise. Sa stricte application s'avérera d'ailleurs parfois impossible dans certaines entreprises, ouvrant le champ de l'interprétation sur le terrain. Enfin, les patrons de PME, de TPE et de commerce sont souvent seuls pour mettre en place ces prescriptions et n'ont donc aucune autre sécurité juridique que celle de leur bon sens. Seuls, ils sont juridiquement

juridique de la reprise d'activité. Il considère que cette inquiétude des chefs d'entreprise peut être légitime et qu'il convient d'y répondre. Vous avez justement rappelé que la nature de l'obligation de sécurité de l'employeur

obligatoires respecte ses obligations légales et peut s'exonérer de sa responsabilité civile.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste et républicain ont déposé plusieurs amendements visant à répondre aux inquiétudes des maires à la suite des décisions et déclarations parfois chaotiques du Gouvernement.

pris en étau entre des injonctions gouvernementales multiples et complexes et une absence criante de moyens et d'accompagnement pour les mettre en oeuvre, s'interrogent sur l'opportunité parce qu'ils sont en première ligne, le risque est réel que pèse sur eux une responsabilité qui ne correspond ni à la part qu'ils ont prise dans la décision ni aux moyens dont ils disposent. Nous considérons que des clarifications et un cadre juridique protecteur sont indispensables. Il est de votre responsabilité de soutenir et d'aider celles et ceux qui ont décidé de vous faire confiance et de vous accompagner dans le déconfinement. C'est pourquoi notre groupe propose que, à compter de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et jusqu'à trois mois après sa cessation, tout acte accompli par un élu local ou un agent public ayant reçu délégation visant à mettre en oeuvre une décision prise par l'État dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire engage exclusivement la responsabilité de l'État. À l'inverse de ce que le Premier ministre a suggéré dans sa déclaration, il ne s'agit pas d'exonérer les acteurs publics de leur responsabilité, mais de situer la responsabilité à son juste niveau. Or en l'espèce, puisque c'est l'État qui décide de tout et tout seul, il ne peut reporter sa responsabilité sur les élus locaux. Ma question est donc simple : le Gouvernement apportera-t-il son soutien à ces amendements ?

dans le cadre du déconfinement ne le fassent pas dans la crainte de voir leur responsabilité pénale engagée. Toutefois, nous le savons aussi, toute décision politique emporte une part de responsabilité qu'il n'est pas question de nier.

pose un cadre très strict qui limite la possibilité d'engager la responsabilité des employeurs publics pour mise en danger de la vie d'autrui ou bien pour des infractions involontaires.

La responsabilité pénale ne peut alors être recherchée que dans deux hypothèses : soit sur la base d'une faute délibérée, c'est-à-dire de la violation délibérée d'une norme existante qui impose une obligation particulière, soit, en l'absence de norme, sur la base d'une faute caractérisée.

la Cour de cassation exige une appréciation de cette éventuelle faute. Au regard de ce cadre juridique, il me semble donc difficile que les élus locaux ou les employeurs qui donneraient les instructions nécessaires en matière de dispositifs liés à la sécurité sanitaire puissent voir leur responsabilité engagée. Nous apprécierons toutefois ensemble si une codification ou une clarification de ces dispositions peut apporter un élément de réassurance supplémentaire. Nous serons prêts à accompagner les travaux du Parlement en ce sens. Madame la garde des sceaux, le Premier ministre a demandé de l'adhésion au processus de déconfinement. En contrepartie de cette adhésion, il vous faut lever les doutes sur la responsabilité. Ces doutes remontent de partout sur le terrain, au sujet des écoles de campagne dont les locaux sont exigus et qui n'ont pas de salle supplémentaire pour faire manger les enfants,

ce service public facultatif. Ce ne sont pas les décrocheurs qui seront les plus volontaires, mais ceux des classes à examen- terminale, première, troisième. Je le regrette. Les conditions dans lesquelles se fera la réouverture des écoles sont un enjeu de taille pour la santé des élèves et de leurs familles, d'autant que le conseil scientifique et le conseil de l'ordre des médecins ne sont pas favorables à leur réouverture. Vous avez pris vos responsabilités ou, plus exactement, vous demandez aux maires d'assurer cette responsabilité en leur laissant ce grand pouvoir de décision : ouvrir leurs écoles

comment les maires pourront-ils garantir qu'une distanciation d'un mètre est assurée dans la cour de récréation, dans les couloirs, dans les sanitaires ? C'est pourtant une indication qui les engage et que vous avez inscrite dans le protocole. Plus il y a de normes, puis il y a de risques de voir un parent d'élève dont l'enfant sera infecté par le Covid-19 saisir les tribunaux et faire inculper ainsi nos élus. Monsieur le Premier ministre, il n'est pas possible de laisser les maires seuls face à ce risque. Ils ont montré leur totale implication pour être à vos côtés dans cette crise sanitaire sans précédent. Ne décidez pas avant la concertation. Nous devons les rassurer, les protéger. Dans le futur projet de loi, aucune disposition ne permet de clarifier les responsabilités des élus dans cette période si singulière. Je vous ai entendu, monsieur le Premier ministre. Nous vous avons senti ouvert à la discussion. J'espère que vous ferez un accueil favorable aux propositions du président de la pour protéger nos élus locaux corvéables à merci, car le déconfinement, c'est demain, et nous ne pouvons pas attendre. La

quel qu'il soit, permette d'empêcher des procédures pénales. Quelle que soit la précision de la loi, il se trouvera toujours un administré ou quelqu'un d'autre pour engager une procédure qui entraînera des jugements. Il faut avoir cela en tête.

Mais si cette échéance nous semble si lointaine, c'est aussi parce que les interrogations sur la levée du confinement, notamment s'agissant des transports, sont encore trop nombreuses. Sommes-nous prêts, monsieur le secrétaire

Dans un courrier du 30 avril, nous apprenions que les principaux opérateurs de mobilité- SNCF, RATP, Keolis, Transdev, pour ne citer que ces derniers -vous informaient que le respect des règles de distanciation physique d'un mètre entre passagers n'était pas réalisable. Pour faire simple, le respect des règles de distanciation veut que le nombre d'usagers dans les transports en commun soit compris entre 10 % et 20 % de la normale. Lundi prochain, il sera de 30 %. Comment allez-vous procéder pour assurer le respect des règles de distanciation ? Vous prévoyez aussi que les masques seront obligatoires dans les transports en commun, et vous avez raison. Néanmoins, comment allez-vous contrôler l'effectivité de cette mesure ? Vous avez précisé qu'il serait possible de réaliser des contrôles grâce aux forces de l'ordre et aux opérateurs de sûreté. Concrètement, quelle sera votre méthode ou stratégie pour que la mesure soit pleinement appliquée ? Mais surtout, en l'absence d'agents pour réaliser les contrôles, un chauffeur de bus, par exemple, pourra-t-il refuser l'accès de son véhicule à une personne sans masque ? Vous avez semblé hésitant à ce sujet dans une précédente intervention. Enfin, quel est votre plan pour distribuer les masques promis il y a encore quelques jours ? La

sécurité sanitaire des voyageurs qui prévaut. je peine à comprendre que les principaux opérateurs de notre pays, dont l'actionnariat est plutôt public, soient obligés de vous envoyer un courrier le 30 avril pour vous demander les modalités de déconfinement au 11 mai. Ces opérateurs publics indiquent qu'il faut 100

indices ou sous-indicateurs : l'indicateur principal- le pourcentage de patients admis aux urgences dans un département donné en lien avec une suspicion de coronavirus -et ce que l'on appelle des signaux faibles- le recours aux médecins généralistes, les remontées des réseaux sentinelles, le nombre d'admissions en réanimation, le nombre de tests positifs réalisés par département.

parfois à l'étranger. Ce bloc régional de saturation des services de réanimation est celui dont nous devons tenir compte pour déterminer si, oui ou non, un territoire est prêt à être déconfiné dans les mêmes conditions qu'un territoire avec peu de malades à l'hôpital et peu de circulation virale. Enfin se pose la question de l'adaptation et de la capacité de réaction de notre système en tests, en traçages

À la demande du Gouvernement, le Sénat est appelé à se prononcer par un vote sur la déclaration du Gouvernement relative à

les secrétaires Catherine Deroche et Agnès Canayer superviseront depuis leur place le déroulement du scrutin.

Le scrutin est ouvert.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure

bien ! D'ailleurs, voilà quelques dizaines de minutes, au moment où nous étions en train de débattre, le Président de la République, de manière spontanée, faisait une conférence de presse sur le déconfinement. J'espère que ses propos étaient conformes à ceux du Premier ministre- et réciproquement.

Dont acte. L'urgence, nous la partageons. En revanche, nous condamnons le fait que le Gouvernement fasse porter à d'autres ses propres difficultés. Vous connaissez l'adage latin : « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

mais la démocratie parlementaire nous incite à reprendre maintenant nos droits- permettez-moi cette expression -et le Gouvernement doit rapidement inscrire à l'ordre du jour des assemblées l'examen des projets de loi de ratification. si le Parlement a autorisé le Gouvernement à intervenir dans des domaines qui relèvent de la loi, c'est à lui qu'il appartient d'avoir le dernier mot. Monsieur le ministre, je vous remercie de prendre en considération ces remarques, qui ont pour but non pas de bloquer votre travail, mais de faire mais de faire respecter le Parlement, en particulier la Haute Assemblée, qui a toujours été constructive dans ses remarques, ses approches et ses préconisations, pour que la crise soit la moins longue possible dans notre pays.

sont un frein à l'utilisation de notre droit d'amendement, qui est un droit constitutionnel. La démocratie parlementaire est bafouée, pour ne pas dire méprisée. Cependant, comme nous sommes des hommes et des femmes politiques très responsables, nous avons

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis un mois et demi, notre pays fait face à l'impensable.

Affronter une crise sanitaire de l'envergure de celle provoquée par le Covid-19 était devenu un impensé, l'impensé d'un monde où le progrès technique et technologique nous protégeait de bien des périls, d'un monde où le sens collectif du tragique avait presque entièrement disparu. Pourtant, en seulement quelques semaines, ce monde a trébuché, faisant trébucher avec lui bien des dogmes et des certitudes. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit confinée. Partout dans le monde, c'est l'appel à rester chez soi qui a été lancé. Rester chez soi, limiter ses déplacements, renoncer à voir des parents ou des amis : autant de sacrifices consentis pour freiner la propagation du virus et protéger les plus fragiles. Avant toute chose, je veux évidemment saluer les soignants, dont chacun mesure l'engagement et qui, chaque jour, se démènent au péril, parfois même au prix de leur vie. La Nation tout entière les regarde avec fierté, parce que rien n'est plus beau que de consacrer sa vie à sauver celle des autres. Je salue de la même manière toutes celles et tous ceux qui permettent à la France de tenir bon et de surmonter cette épreuve. Grâce à eux, notre pays n'a pas sombré dans le chaos,

a poursuivi son activité, parce que, même quand la vie du pays semble s'arrêter, la démocratie, elle, ne s'arrête jamais. J'entends vos critiques sur les jamais. J'entends vos critiques sur les délais extrêmement contraints dans lesquels vous avez été amenés à examiner le projet de loi que je vous présente aujourd'hui. Bien sûr, nous aurions souhaité que vous disposiez de davantage de temps. Bien sûr, nous respectons la vie démocratique et la vie parlementaire de ce pays. C'est pourquoi, semaine après semaine, le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont présents dans cet hémicycle, comme à l'Assemblée nationale : la continuité du fonctionnement de nos institutions

Je salue aussi, à travers vous, l'engagement remarquable des élus locaux, qui, dans tous les territoires, ont pris des initiatives, ont inventé et ont joué un rôle décisif dans la protection des populations. Le quotidien de notre pays a été bouleversé. Il le fallait pour éviter le pire. Nul ne peut s'en réjouir et tout le monde s'en serait volontiers passé. Les décisions prises jusqu'à présent dans ce contexte n'ont rien d'anodin et le Gouvernement en a parfaitement conscience. Le Gouvernement sait que le texte qui vous est proposé et qui est destiné à proroger l'état d'urgence sanitaire n'est pas un blanc-seing. Bien au contraire, le Gouvernement mesure la responsabilité immense, la responsabilité historique qui est la sienne aujourd'hui. L'état d'urgence sanitaire n'a qu'une seule vocation : permettre la lutte la plus rapide et la plus efficace possible contre l'épidémie qui frappe. Ce projet de loi visant à proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet prochain est, conformément à l'avis unanime du comité de scientifiques, une nécessité. à l'unanimité, le conseil scientifique a considéré que l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'épidémie de Covid-19 incluant ceux qui ont été prévus par la loi sur l'état d'urgence sanitaire restent nécessaires dans la situation sanitaire actuelle et pour les semaines, voire les mois à venir. Je profite de mon intervention pour vous donner l'état des lieux aujourd'hui dans notre pays vis-à-vis de l'épidémie ; chacun pourra ainsi se rendre compte de la situation à laquelle nous faisons face. Ce soir, 131 863 patients ont été diagnostiqués et confirmés par test PCR pour le coronavirus ; ce sont 576 patients de plus au cours des vingt-quatre dernières heures.

il y a une situation hospitalière qui reste tendue, difficile ; il y a une épidémie que nous avons combattue avec succès grâce au confinement et grâce à l'action des Français depuis de nombreuses semaines, mais que nous n'avons pas totalement vaincue, tant s'en faut. C'est pourquoi le Gouvernement sollicite la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Il a aussi semblé que, après six semaines au cours desquelles le pays tout entier a appris à vivre autrement, il convenait de proposer quelques modifications ciblées du régime de l'état d'urgence sanitaire afin d'en conforter le cadre juridique. Je l'ai dit à Philippe Bas, président de la

de pouvoir débattre avec vous afin que nous puissions avancer ensemble pour enrichir ce texte, le consolider et le conforter partout où cela sera nécessaire. C'est surtout la perspective du déconfinement qui a amené à accélérer l'examen de ce projet de loi, compte tenu des adaptations législatives qu'il implique, et à prévoir un examen parlementaire compatible avec une entrée en vigueur du déconfinement le 11 mai Le déconfinement qui s'opérera peu à peu à partir de cette date ne sera pas un retour pur, simple et immédiat à la vie d'avant ; le Premier ministre l'a dit : il va falloir vivre avec le virus.

J'ai souvent comparé ce que nous vivions à une course de fond : le 11 mai correspondra au premier ravitaillement de cette course de fond, mais le chemin sera encore long avant de franchir la ligne d'arrivée. Des vies sont en jeu ; la bataille n'est pas encore gagnée, loin de là. de le dire, il est indispensable de sécuriser et d'élargir le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire afin d'y intégrer les enjeux du déconfinement. Je pense en particulier à la réglementation dans les transports ou les établissements recevant du public.

Le projet de loi permet de mieux encadrer les possibilités de placement en quarantaine ou à l'isolement. Il renforce les garanties, notamment juridictionnelles, qui s'y rapportent. Les conditions générales seront définies par décret, après avis du comité de scientifiques. Je pense en particulier à la durée de ces mesures, aux lieux dans lesquelles elles pourront s'appliquer, au suivi médical qui les accompagnera, ainsi qu'aux déplacements que les personnes concernées pourront, le cas échéant, effectuer ou, à défaut, les moyens par lesquels un accès aux biens et services de première nécessité leur sera garanti. J'y insiste, les mesures individuelles prises sur ce fondement ne pourront viser que ceux qui entrent sur le territoire national ou qui arrivent dans un territoire ultramarin ou en Corse, ou en provenance de l'un de ces territoires. Le Gouvernement n'a pas retenu la possibilité d'appliquer ces mesures aux personnes affectées par le Covid-19 qui auraient refusé de manière réitérée des prescriptions médicales prophylactiques et créeraient par leur comportement un risque de contamination pour d'autres personnes. Notre volonté, comme j'ai eu l'occasion de le dire au président Milon, est avant tout de faire confiance et de responsabiliser. Les mesures individuelles seront prononcées sur décision motivée du représentant de l'État, sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé et sur constatation médicale de l'infection en cas de placement à l'isolement. Bien évidemment, et c'est heureux, les mesures individuelles interdisant toute sortie

J'ai noté avec satisfaction que la commission des lois a souhaité apporter un certain nombre de garanties, de précisions, dont nous pourrons débattre dans quelques minutes. Enfin, les mesures en cause ne pourront en aucun cas se prolonger au-delà de trente jours.

Tout ce qui peut aider à lutter contre ce virus doit être exploité, pas n'importe comment, bien sûr, mais en veillant scrupuleusement au respect des principes auxquels nous sommes toutes et tous attachés. J'y reviendrai. reviendrai. Avec ce système d'information, il s'agit de collecter un grand nombre de données d'ordre médical et non médical pour les porter à la connaissance de différents intervenants, avec cinq étapes distinctes.

pour enrichir la liste des cas contacts au-delà de ce premier cercle et vérifier qu'aucun cas positif n'a échappé au de niveau 1 avant de donner toutes les consignes aux intéressés.

vise à diligenter les enquêtes de terrain là où il y a une circulation encore plus active et concentrée du virus sur un territoire donné, de manière à casser, à briser les chaînes de contamination et à éviter des flambées épidémiques. Enfin, cinquième étape : la surveillance épidémiologique locale et nationale effectuée par Santé publique France et la direction générale de la santé. Je veux être très clair : ce système d'information est destiné à identifier des personnes infectées ou susceptibles de l'être, à collecter des informations nécessaires pour déterminer les personnes ayant été en contact avec ces dernières, à organiser des examens de biologie médicale de dépistage et à réaliser toutes choses utiles dans la lutte contre la propagation du virus.

Ces systèmes d'information existent depuis des années et même des décennies. Y ont accès aussi bien des médecins, des pharmaciens que des salariés de l'assurance maladie, qui ne sont pas forcément médecins.

Comme il n'a jamais été envisagé de donner accès aux mêmes acteurs de l'assurance maladie, aux mêmes médecins, aux mêmes soignants à des fichiers de personnes qui ne sont pas forcément malades, nous avons besoin de recourir à la loi. C'est tout l'intérêt de cette disposition législative. Je veux aussi couper court à toute suspicion et à toute polémique. Les données concernées ne seront pas récoltées pour nourrir une application. Les systèmes d'information dont nous parlons sont juridiquement et techniquement

d'avoir accès à un seul système d'information où vont pouvoir interagir des médecins, des infirmiers, des biologistes et des salariés de l'assurance maladie. La mise en oeuvre de ces mesures supposera un décret en Conseil d'État, pris après un avis de la CNIL, qui sera rendu public, et qui est d'ores en préparation. Mesdames, messieurs les sénateurs, je n'ai pas manqué de saluer voilà quelques instants, à travers vous, tous les élus locaux de notre pays. Si l'on peut trouver une seule vertu à la crise sans précédent que nous traversons, c'est bien de révéler l'engagement et le sens des responsabilités des uns et des autres ; c'est de mettre à l'épreuve un système de décision en le confrontant à ses atouts, certains, comme à ses limites, tout aussi certaines. tout aussi certaines. Personne n'oubliera que, face au péril, les élus locaux, qu'ils soient maires, élus régionaux ou départementaux, ont été pleinement mobilisés pour organiser le combat contre le virus. Je pourrais en dresser la liste,

La période de déconfinement qui s'annonce verra les territoires jouer encore, forcément, un rôle très actif. Le texte que le Gouvernement présente aujourd'hui est équilibré, gage d'efficacité dans le combat contre le virus, respectueux de principes avec lesquels nous ne transigerons jamais.

de tous. La parole est à M. le rapporteur. Monsieur le ministre, je n'ai pas besoin de vous le dire, car vous le savez déjà, le Sénat tout entier est mobilisé pour participer à la lutte contre ce fléau épouvantable qu'est ce nouveau coronavirus, qui donne la maladie dite du Covid-19. Nous le sommes avec le souci de ne prendre des mesures contraignantes pour nos concitoyens que lorsqu'elles sont strictement nécessaires, en préservant toujours, autant qu'il est possible dans cette période exceptionnelle, nos libertés, nos droits fondamentaux et la vie privée. Il est d'ailleurs très difficile de trouver le bon point d'équilibre, et je ne suis pas sûr que nous y parviendrons. D'une certaine façon, je pense que la vigilance du Conseil constitutionnel permettrait de prendre le relais de la nôtre. Il me paraît tout à fait important que nos concitoyens sachent que, si nous menons avec résolution ce combat, nous avons l'exigence de lutter avec les armes qui sont celles d'une grande démocratie et d'un État de droit.

le moyen de s'exprimer davantage devant les Français, même s'il reste, de notre point de vue, un certain nombre de zones d'ombre entourant la journée du lundi 11 mai. Monsieur le ministre, vous nous présentez aujourd'hui ce texte.

Gouvernement. Il comporte des mesures certes importantes, mais elles sont ponctuelles. J'ai proposé à la commission des lois de les adopter, moyennant un grand nombre de modifications, dont certaines, très importantes, nous ont été inspirées par la commission des affaires sociales. Le président Milon s'exprimera dans un instant sur ces propositions. Ce texte comporte- dans la mesure où nous sommes dans la discussion générale, je vais me cantonner aux généralités

Nous avons inscrit des garanties supplémentaires. Je rappelle que c'est surtout pour les outre-mer que vous avez besoin de ces mesures de quarantaine, même si elles peuvent s'appliquer à d'autres circonstances lors de l'entrée sur le territoire national. Nos îles

il y a des mesures qui relèvent du système d'information que vous voulez mettre en place. Ne nous arrêtons pas trop sur le système d'information, car, ce qui est important, c'est ce que vous voulez en faire. Nous sommes majoritairement d'accord avec la finalité que vous avez retenue. Quelle est-elle ? Il s'agit de remonter les filières de contamination. À un malade ou à quelqu'un qui s'est révélé porteur du virus,

d'accepter de se mettre en quatorzaine pour ne pas courir le risque de contaminer autrui. Nos compatriotes, qui sont de bons citoyens- ils l'ont prouvé pendant le confinement

nous avons accepté en commission des lois de le mettre en place, mais à une condition majeure : le Gouvernement doit accepter un certain nombre de garanties supplémentaires, sur le détail desquelles je ne m'attarde pas maintenant, car nous aurons largement le temps de le faire tout à l'heure.

finalement, le confinement est plus facile que le déconfinement. Le confinement, c'est une règle applicable à tous, sur tout le territoire national : vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, sauf

c'est une multitude de situations qu'il va falloir régir : dans les transports, dans les écoles, dans les entreprises, dans les administrations et même dans les rues.

il est également important que les masques soient accessibles aussi massivement que possible. D'ailleurs, spontanément, les Français veulent en porter. Vous pouvez le vérifier tous les jours. Par ailleurs, nous avons besoin

Ainsi, au moment du déconfinement, ce n'est plus l'État qui va dire : « À mes ordres, adoptez le comportement de confinement ! Ce sont des dizaines de milliers de personnes, qui, chaque jour, vont prendre des décisions. Parmi elles, il y aura des maires, des présidents de grandes collectivités et leurs collaborateurs ; il y aura aussi des chefs d'entreprise. vont prendre des risques dans l'organisation du travail ; elles vont prendre des risques pour le bon accueil des enfants à l'école. Nous voulons permettre à ces décideurs de prendre ces risques sans s'exposer

non seulement pour vous demander de revenir nous voir plus tôt que vous ne l'aviez prévu si vous voulez prolonger l'état d'urgence, mais aussi pour exiger un aménagement temporaire de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de tous ceux qui vont avoir à prendre des risques raisonnés pour permettre au déconfinement progressif de réussir.

depuis l'adoption de la première loi d'urgence, je ne peux entamer mon propos sans vous faire part d'une grande satisfaction, dont la période qui s'achève s'est pourtant montrée particulièrement avare pendant que le pays, dépourvu à ce jour de toute certitude sur son avenir, est engagé dans un moment de son histoire dont il gardera pour longtemps la mémoire et les marques, le Parlement, en particulier le Sénat, n'a pas un instant cessé d'exercer, dans la tempête sanitaire qui nous secoue violemment, la vigilance essentielle et indispensable à tout état d'exception. Sur le texte soumis aujourd'hui à notre examen, par lequel le Gouvernement nous demande de proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet, la commission des affaires sociales s'est saisie pour avis de trois articles et a adopté six amendements, dont cinq ont été retenus par la commission des lois. Un point divise donc nos deux commissions. À mon sens, il résume à lui seul les conditions de la réussite que l'on est en droit, non pas seulement d'espérer, mais d'exiger de la levée du confinement. Lors de sa déclaration devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a érigé le point saillant de sa stratégie en un triptyque, dont la célébrité a presque immédiatement concurrencé celle de notre devise républicaine : protéger, tester isoler des mots vibrant et généreux, dont le succès ne pourra cependant dépendre d'une simple incantation. Après la levée progressive du confinement, dont on ne peut qu'accueillir la nouvelle avec soulagement, monsieur le ministre, faire supporter la lutte contre l'épidémie, fort loin d'être remportée, sur la seule responsabilisation citoyenne des personnes, y compris celles qui continueront d'être atteintes par le virus et celles qui, par leurs contacts, seront susceptibles de l'être. J'entends bien l'obligation politique d'emprunter désormais des voies décisionnelles, qui, après deux mois d'enfermement imposé à nos concitoyens, privilégient l'incitation à la contrainte. Les professionnels de santé auditionnés par la commission des affaires sociales et engagés dans les premières formes de suivi sanitaire à domicile des patients atteints nous ont rappelé cette condition première et fondamentale, que vous connaissez en tant que praticien, et à laquelle tout soignant se doit de toujours soumettre son action : le consentement et l'adhésion de son patient. Je ne souhaite pas, bien évidemment, remettre en cause ce principe, mais que sait-on vraiment, mes chers collègues, de l'horizon maintenant tout proche que la levée du confinement dessine ? Victimes de l'enthousiasme bien légitime qui nous prend au moment où nous annonçons à nos concitoyens que leur liberté d'aller et venir sera bientôt recouvrée, n'oublierions-nous pas un peu vite que le matin du 11 mai ne rangera pas magiquement les ravages de cette épidémie dans les épisodes malheureux, mais clos, de notre histoire Le risque d'un sursaut de la maladie, avec la cohorte tragique d'hospitalisations qui l'a accompagnée, est aussi réel et présent qu'à ses premiers jours. La seule différence entre hier et aujourd'hui tient dans la capacité de notre système hospitalier, qui, exemplaire dans la prise en charge de la première vague, ne manquerait pas d'être irrémédiablement submergé par la seconde. Inciter à un changement réel des comportements individuels est nécessaire, mais quel poids accorder au premier mot lancé par le Premier ministre- « protéger » -si on lui refuse l'appui du troisième, à savoir « isoler » ? Le texte du Gouvernement réserve les quarantaines et isolements aux seuls mouvements de population transfrontaliers ou interinsulaires. Ce n'est pas seulement insuffisant, n'est pas seulement insuffisant, c'est dangereux. Par cette qualification des seuls cas d'isolement prophylactique contraint, monsieur le ministre, vous faites courir à nos concitoyens le risque d'une insouciance périlleuse, qui considérerait le danger écarté tant que l'on reste à l'intérieur de nos frontières. L'histoire nous prouve que ces craintes ne sont pas infondées et que les appels les plus renouvelés à la responsabilité citoyenne peuvent se montrer cruellement insuffisants. Les épidémiologistes ont tous en mémoire

À ceux qui me rappelleront justement que l'on ne pourra pas reconstruire notre société et notre économie durement éprouvées en substituant la diffusion du soupçon à celle du virus, je répondrai que la confiance ne se conçoit pas sans précaution.

démocratique face à la violence de l'épidémie, qui peut expliquer la légèreté du contrôle de constitutionnalité sur des dispositions particulièrement lourdes en matière de libertés publiques et démocratiques. La précipitation exigée par cette agression virale, mais aussi par un état d'impréparation de dénuement de notre pays face à une telle situation, que nos concitoyennes et nos concitoyens ne comprennent toujours pas, a provoqué le transfert d'une forme de pleins pouvoirs au Gouvernement pour une durée indéterminée. Il est grand temps de vérifier si l'état d'urgence que nous vivons et sa prolongation sont conformes à la Constitution et aux valeurs fondamentales de notre République. Cela ne fait pas de doute, ce projet de loi sera soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel, et nous nous associons à cette démarche. Il nous paraît cependant nécessaire que le Parlement, notamment le Sénat, débatte dès maintenant de cette constitutionnalité, exerçant ainsi son pouvoir souverain, sans attendre l'examen par le Conseil constitutionnel, lequel, dois-je le rappeler, n'est pas pourvu de la même légitimité démocratique et a pris une décision contestable et contestée sur la loi organique du 25 mars dernier accompagnant le premier état d'urgence sanitaire. Depuis le 16 mars, notre pays est confiné. Les libertés publiques et la démocratie le sont aussi. Le Gouvernement et son administration ont pris seuls les rênes du pouvoir : ont été pris 31 ordonnances, 70 décrets, autant d'arrêtés ministériels et au moins 1 200 arrêtés préfectoraux. Action Action et efficacité ont été les maîtres mots du Président de la République, de son Premier ministre et des ministres. Bien sûr, il fallait agir vite ; bien que la mobilisation soit générale et exemplaire. Toutefois, monsieur le ministre, nous constatons que cette prise en main de la quasi-totalité des pouvoirs s'est traduite par une forme d'infantilisation de notre peuple et de ses représentants. « Ayez confiance », clamez-vous à tout-va. Mais, en démocratie,

à l'écoute de ses difficultés, de ses souffrances, de ses inquiétudes, de ses colères et de ses exigences. Le Président de la République a admis des failles, des lenteurs, des insuffisances. C'est plutôt, selon nous, la faillite d'un système libéral fondé sur la réduction d'une dépense publique entraînant la casse des services publics, en premier lieu lieu de l'hôpital, qu'il faut admettre une fois pour toutes. Le triste feuilleton des masques et la longue incapacité de production de tests le soulignent : les pleins pouvoirs ne résolvent pas tout. tout. Le temps perdu par des choix politiques et non pas par la fatalité ne se rattrape pas par une débauche de communication souvent désordonnée et contradictoire, mais par une mobilisation de tous les acteurs de notre démocratie : les citoyennes et citoyens, les forces associatives et syndicales, les parlementaires, les élus locaux et l'exécutif. Comment ne pas constater que la captation de tous les pouvoirs par ce dernier est d'autant plus insupportable démocratiquement que notre pays est confronté depuis des années à une centralisation des décisions aux mains

aurait dû être préalablement débattue, partagée, sous-pesée par les acteurs démocratiques, économiques et sociaux. Tel n'a pas été le cas, puisque de nombreux membres du Gouvernement ont eux-mêmes découvert cette décision au dernier moment.

d'amendement et de vote. Faute de masques, faute de tests, faute de préparation dans les transports, faute de moyens, la date du 11 mai devient incertaine, et ce qui aurait dû être source d'espoir est devenu source de profonde inquiétude. La situation de défiance qui monte dans notre pays indique qu'il faut maintenant restaurer le fonctionnement démocratique de nos institutions. La question de la levée de l'état d'urgence est donc posée. Cet état d'urgence est

un nouvel état de crise : l'état d'urgence sanitaire. Il y est précisé que la prorogation de l'état d'urgence au-delà d'un mois doit être autorisée par la loi. Il y est aussi précisé que la loi, confirmant cette prorogation d'un mois, doit en fixer la date butoir. effet, le nouvel article L. 3131-14 du code de la santé publique dispose : « La loi autorisant la prorogation au-delà d'un mois de l'état d'urgence sanitaire fixe sa durée.

Le troisième alinéa de l'article 4 indique en effet que la prorogation de l'état d'urgence, le second état d'urgence, à savoir l'exception de l'exception, au-delà de la durée de deux mois ne peut être autorisée que par la loi. Plus d'obligation, donc, dans cette situation, de prévoir une date butoir. Nous contestons la constitutionnalité de cet article 4, lequel, rappelons-le, n'a pas été soumis au Conseil constitutionnel après Monsieur le président de la commission des lois, je sais que la question de la maîtrise par le Parlement de la durée de l'état d'urgence était pour vous une priorité. En 2015, lors de l'examen du projet de révision de la Constitution relatif à la protection de la Nation, qui n'a finalement pas abouti, vous aviez déposé deux amendements significatifs pour préserver le pouvoir pour préserver le pouvoir des assemblées en matière de fixation de la durée de l'état d'urgence. L'un de ces amendements visait même à garantir le le pouvoir des assemblées, y compris dans le cas des articles 16 et 36, relatifs à l'état de siège et aux pleins pouvoirs. Quelle que soit la gravité de la crise, le transfert massif du pouvoir législatif au pouvoir exécutif pour une durée indéterminée n'apparaît pas conforme aux valeurs de la République ni à l'esprit même de la Constitution. Avant tout examen du texte, nous devons demander au Gouvernement de rétablir l'équilibre institutionnel, en fixant une date butoir à l'état d'urgence. En effet, ne l'oublions pas,

retenues. Option 1 : ne pas modifier le cadre législatif en continuant de s'appuyer sur les dispositions sanitaires existantes des articles L. 3131-1 du code de la santé publique et d'autres dispositions plus spécifiques du même code en matière de réquisition ou encore de lutte contre la propagation internationale des maladies, ainsi que sur le pouvoir de police appartenant respectivement au Premier ministre, aux maires et aux préfets. Option 2 : compléter les dispositions existantes pour les adapter aux situations extrêmes. Option 3 : l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit d'une pleinement politique, dont la pertinence sanitaire reste à prouver. Limiter la durée de l'état d'urgence est une exigence constitutionnelle. Le Défenseur des droits a d'ailleurs rappelé « l'impératif de limiter dans le temps les dispositions spéciales qui restreignent l'exercice des libertés publiques ». de proroger l'état d'urgence et non pas de le limiter. Nous refusons clairement cette disposition. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons déposé cette motion tendant à opposer

Cette vision n'est pas la nôtre ! Nous sommes les représentants de la Nation au Parlement, au Sénat de la République, et jamais nous ne pourrons l'accepter. Nous Nous ne sommes pas non plus les apôtres d'un système dans lequel il n'y aurait plus les garanties de l'État de droit pour s'opposer aux excès de pouvoir. Quand nous nous prononçons en faveur de l'état d'urgence sanitaire, cela ne signifie pas que nous renoncions à l'État de droit, car nous prévoyons des garanties.

de véritables sources de préoccupation, que vous avez exprimées et que je partage s'agissant de l'équilibre des pouvoirs dans la République et d'un certain nombre d'évolutions qui ne me paraissent pas favorables à la vie d'une démocratie équilibrée dans laquelle tous les points de vue peuvent être entendus avant la décision. Reste que nous sommes là et que nous ne pouvons pas, sans nier notre propre mission, considérer que le Parlement n'aurait pas d'importance. Nous voterons- ou pas

depuis le début de la crise sanitaire, les élus locaux, les maires et les parlementaires se sont engagés pour appliquer localement la stratégie décidée par le Gouvernement. Nous avons fait preuve de bonne volonté et de bienveillance, car cette crise exige de notre part une implication totale et constructive. constructive. Le projet de loi qui nous est présenté devrait constituer une étape décisive dans le processus de déconfinement, mais il pose plus de questions qu'il n'en résout. Nous en avons tous conscience, le déconfinement est une étape complexe. Les acteurs de terrain, notamment les maires et les chefs d'entreprise, qui seront confrontés à de nombreux défis, sont en première ligne. Pourtant, ce texte ne dit rien sur leurs missions précises et les moyens qui leur seront donnés pour agir. La question de leur responsabilité juridique, qui aurait dû être abordée rapidement, ne trouve toujours pas de réponse. C'est pourtant la base avant leur implication dans une stratégie qui reste floue à bien des égards. Aujourd'hui, la date du déconfinement est encore suspendue à des indicateurs qui sont biaisés, car le confinement seul ne suffit pas. Pour être efficace, il fallait avoir une stratégie globale reposant sur des protections en nombre, des tests de dépistage et une phase d'isolement d'isolement des personnes contaminées. C'est ce qui a été fait dans plusieurs pays, et ce depuis plusieurs semaines. Dans ce projet de loi, de nombreux sujets sont renvoyés à des ordonnances et à des décrets ultérieurs. Ainsi, l'article 3 évoque les plans d'accompagnement, mais ne précise pas le rôle des maires

l'article 6, relatif à l'organisation des systèmes d'information et à la surveillance locale des cas détectés, il ne donne pas non plus les garanties nécessaires ni le cadre légal indispensable sur un sujet aussi sensible. Enfin, la reprise économique constitue un pilier majeur dans le dispositif du déconfinement. Les chefs d'entreprise sont eux aussi en première ligne. Ils ne doivent pas être tenus responsables des risques sanitaires dus au Covid-19. Comme pour les maires, leur faire porter une responsabilité juridique, éventuellement pénale, sans l'avoir définie au préalable est inacceptable. Ces lacunes constitueraient un frein au redémarrage économique du pays, sur lequel repose notre avenir. En conclusion, je tiens à dire que, si je ne m'oppose pas à l'adoption de cette loi, de nombreuses questions restent en suspens.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a six semaines, nous débattions de la mise en oeuvre d'un état d'urgence sanitaire spécifiquement créé pour lutter contre le Covid-19. Notre groupe avait alors émis de nombreux doutes sur ce régime d'exception. Nous avions mis en garde sur l'effacement du contrôle parlementaire et, plus généralement, sur les garanties démocratiques données aux Français et à leurs élus. Aujourd'hui, le déconfinement progressif du pays est envisagé pour le 11 mai dans une grande confusion. le Sénat vient d'émettre un avis défavorable sur le plan de déconfinement du Gouvernement. Le même jour, monsieur le ministre, vous nous demandez de prolonger l'état d'urgence de deux mois et d'en étendre les dispositions, comme si la méthode actuelle ne devait pas être réévaluée et modifiée. Cette loi d'urgence a habilité le Premier ministre, mais aussi les préfets, à prendre des mesures qui touchent en de nombreux domaines à la restriction des droits et libertés individuelles et collectives. Si personne ne réfute l'urgence sanitaire, une telle situation nécessite une grande concertation, laquelle a largement fait défaut, comme on peut le constater pour l'école. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, après avoir mis en place son propre observatoire de l'état d'urgence, s'interroge dans son avis du 28 avril sur la pertinence de la création d'un état d'urgence sanitaire au regard des textes existants, ainsi que sur son impact sur le fonctionnement des institutions et de la vie démocratique. L'expérience de l'état d'urgence prévu par la loi du 3 avril 1955, maintes fois prorogé à la suite des attentats de 2015, a montré que le risque de contamination du droit commun

posent problème. Dans les transports, alors que vous ne répondez ni aux alertes des opérateurs de transport public sur le déconfinement ni à l'appel à un soutien public massif à la SNCF, vous proposez l'extension des pouvoirs de police visant à verbaliser les usagers des transports à tous les agents des transports publics, ce que ne demandent ni les entreprises concernées ni leurs salariés. Les pouvoirs de police doivent rester du domaine des forces de police,

en discussion, la Cour européenne des droits de l'homme considère que la mise en quarantaine doit constituer le moyen de dernier recours pour empêcher la prolongation d'une maladie. Par conséquent, d'autres mesures moins sévères la Cour européenne, avoir déjà été envisagées et jugées insuffisantes. Or, sur ce point, le projet de loi est flou. Il y a donc un risque à envisager de nouvelles mesures coercitives de cette nature, dans le cadre d'un contrôle parlementaire et juridictionnel aussi réduit et mis en oeuvre dans des temps trop limités.

: gratuité des masques dans les transports et prolongation de l'interdiction des expulsions locatives. Enfin, dernière mesure phare proposée par le Gouvernement, la mise en place d'un large système d'information doit contribuer à identifier les chaînes de contamination. Si le texte législatif évoque ce point, que le dispositif proposé oblige notamment- malgré vos explications, monsieur le ministre -à lever le secret médical, en autorisant l'accès à des données médicales par des personnes non médecins. Les commissions des lois et des affaires sociales ont souhaité apporter plusieurs garanties, selon nous, cela reste insuffisant. La notion de recueil volontaire des données ne figure pas dans le projet de loi et l'anonymat n'est pas garanti. globalement, sur cet article 6, il ne nous paraît pas acceptable de proposer au législateur d'adopter un dispositif aussi important et aussi flou, en laissant aux décrets d'application toute latitude quant au champ précis du système et à sa mise en oeuvre.

En revanche, la déresponsabilisation des chefs d'entreprise, que certains veulent mettre en parallèle, n'est pas acceptable. Toute entreprise se doit de mettre en oeuvre les conditions suffisantes pour assurer la sécurité de ses employés. Après les entorses et les dérogations déjà apportées au droit du travail par l'état d'urgence, de telles mesures ouvriraient la porte à tous les abus, pour pousser au retour au travail dans n'importe quelles conditions. Voilà pourquoi c'est en toute responsabilité que nous voterons contre ce projet de loi.

monsieur le ministre, mes chers collègues, la pandémie du coronavirus a bouleversé le monde. Elle a atteint nombre de nos concitoyens et mis notre pays à l'arrêt. Cette situation sanitaire inédite constitue un défi majeur, en nous imposant de modifier nos comportements au nom de l'intérêt général. Le civisme est une arme primordiale dans le combat qui est engagé. Pour endiguer le virus, des mesures de confinement ont été prises : il a fallu réduire les contacts et les déplacements au minimum. Je tiens tout particulièrement à saluer policiers et gendarmes, qui ont veillé et continuent de veiller au bon respect des mesures de confinement. À cet égard, il est incompréhensible qu'ils ne disposent pas toujours de protection. Je veux saluer aussi les maires, les élus locaux et l'ensemble des collectivités locales, qui se sont montrés à la hauteur de la situation. Le projet de loi que nous allons examiner doit proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au mois de juillet. Ce texte traite de la mise en quarantaine, de l'isolement des personnes infectées et de la collecte des données médicales pour remonter et casser les chaînes de transmission du virus. À titre personnel, je serai vigilant s'agissant de la configuration du dispositif de traçage numérique envisagé par le Gouvernement et visant à informer l'utilisateur de son exposition à un risque particulier de contamination, du fait des personnes rencontrées. Je serai également attentif aux moyens humains déployés qui composeront les brigades d'enquêteurs au niveau territorial. Avant de conclure, je souhaite exprimer ma reconnaissance à celles et ceux qui donnent toute leur énergie pour assurer les soins médicaux et la continuité des activités essentielles. Je veux aussi faire part de ma compassion à tous ceux qui ont perdu un être cher et n'ont pas pu l'accompagner dans leurs derniers instants. Monsieur le ministre, nous devons réussir ensemble le déconfinement. La confiance est l'une des conditions essentielles et majeures pour réussir cette sortie de crise.

qui concerne les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner. Ces ressources des départements sont déjà dans le rouge. Il faut aussi redonner au maire le pouvoir de signer des permis de construire. L'administration devra retrouver son plein niveau afin de combler les nombreux retards qui se sont accumulés. Elle devra être aux côtés de nos concitoyens dans la reprise qui s'amorcera lundi prochain. Le groupe Les Indépendants soutient les orientations de ce projet de loi. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les élus du groupe centriste abordent ce texte dans

que le Parlement donne à l'exécutif les moyens de faire face à une situation de crise extrêmement lourde.

oui au partage d'information au stade de l'enquête épidémiologique de terrain, mais non à cette identification dans des serveurs centraux, qui- je le dis sans aucune discourtoisie à votre égard : c'est le principe qui est en cause -sont à la main du ministère

la première, qui va saisir les résultats dans le système ? Au sujet de la deuxième, comment allez-vous garantir l'anonymat des personnes atteintes par le virus lorsque la chaîne des contacts sera remontée et que les gens seront interrogés ?

En troisième lieu, la crédibilité de ce texte dépend des capacités de fourniture, dans un contexte cohérent,

Or nous ne pourrons pas discuter de toutes les questions sociales, qu'abordera ma collègue Laurence Rossignol, ainsi que de nombreux sujets comme le logement, les centres de rétention,

je n'ai pas besoin de rappeler les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, ni de mentionner le nombre de victimes du Covid-19 en France et dans le monde. Mes toutes premières pensées s'adressent à elles et à leurs familles. Elles vont ensuite à toutes les personnes qui, au sein du corps médical et au-delà, dans ce qu'on appelle désormais les services essentiels, ou encore par un mouvement de solidarité spontanée, ont fait et font tenir notre pays aujourd'hui. J'y reviendrai.

je tiens à saluer la mobilisation qui s'est manifestée sur toutes les travées, pour faire vivre le débat parlementaire malgré les délais particulièrement courts qui nous sont imposés et, en amont, permettre le suivi des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le président de notre groupe, Jean-Claude Requier, l'a déjà indiqué, les membres du RDSE soutiennent la volonté du Gouvernement d'engager la phase de déconfinement. Cependant, nous aurions souhaité que la prorogation de l'état d'urgence comporte des prémices législatives d'adaptation structurelle de notre pays

Je pense bien sûr à l'adaptation de notre système de santé. De façon plus prospective, se posera également la question de l'indépendance alimentaire, que nous avions d'ailleurs soulevée avec la proposition de résolution de Françoise Laborde, l'indépendance pharmaceutique, au moins au niveau européen, ou encore de l'adaptation de l'aménagement du territoire : cette crise a montré à la fois les limites d'une économie dominée par des métropoles extrêmement denses et les vertus de la proximité.

d'autant que la première phase de l'état d'urgence court jusqu'au 23 mai- il s'agissait déjà d'un délai dérogatoire par rapport au régime de droit commun. Où était l'urgence ? Comment évaluer l'impact des mesures proposées sur les personnes chargées de les appliquer sans disposer du temps nécessaire pour les auditionner ? de M. le rapporteur, la majorité des membres du groupe du RDSE n'est pas favorable au fait d'étendre le délai de prorogation au-delà de deux mois, compte tenu des mesures liberticides prévues par ce régime exceptionnel destiné à affronter l'urgence.

de la commission. Ce matin encore, après une analyse de quelques jours, ou plutôt de quelques heures, ce texte faisait naître plus de questions qu'il n'apportait de réponses, même si nos échanges en commission des lois ont permis de lever quelques incompréhensions.

seront les personnes habilitées à recueillir les données médicales dont il s'agit ? à quelle fin ? au moyen de quel support électronique ? au moyen d'un énième système d'information, comme le prévoit l'article 6 ? N'oublions pas que ces personnes manipuleront, principalement, des données personnelles et médicales.

Nous craignons que nos ressortissants des outre-mer passant par des zones de transit y soient soumis ; en résulterait une rupture de la continuité territoriale. Dans certains cas, ces zones de transit sont un passage obligé- je ne citerai que l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon, que nous a rappelé notre collègue Stéphane Artano. Pour le moment, le virus n'a pas disparu, mais nous apprenons à vivre avec lui. Cela implique de retisser le lien de confiance entre nos concitoyens, que les distanciations sociales fragilisent immanquablement. nous disposons de deux ressorts efficaces. Le premier, c'est l'exemple des gestes de solidarité que nous avons observés dans les moments les plus durs du confinement : une grande solidarité s'est manifestée en faveur des travailleurs essentiels, par des actions individuelles ou collectives, notamment associatives, par des actions symboliques ou concrètes. c'est l'espoir de développer des solutions médicales pour lutter contre le Covid-19 à tous les stades de la maladie : les tests, les vaccins ou encore les traitements destinés à limiter les symptômes.

au succès futur de nos enfants et à l'équilibre des familles. Bien sûr, ce travail pose la question de l'élargissement de la protection de nos collègues élus locaux et des autres responsables publics, étant donné la responsabilité légale qu'ils engagent par leurs actes.

tout d'abord, au nom du groupe Les Républicains, je salue l'engagement et le courage des professionnels de santé et je rends hommage à l'ensemble des salariés et des fonctionnaires qui assurent le maintien des services essentiels à la population depuis le début de la crise. Les circonstances exceptionnelles qui nous réunissent appellent, certes, des mesures exceptionnelles, mais les conditions d'examen qui nous sont imposées pour ce texte ne sont pas propices au travail du Parlement. Depuis le vote de la première loi d'urgence sanitaire, plus de six semaines se sont écoulées. Or nous travaillons aujourd'hui sur un texte dont le contenu est connu depuis seulement quarante-huit heures et dont l'examen en commission a eu lieu ce matin même. Le Gouvernement aurait très bien pu organiser la présentation de ce texte dans des délais moins contraints. J'en viens au texte. L'ensemble des mesures de ce projet de loi ainsi que leurs enjeux ont été parfaitement présentés par les présidents-rapporteurs Philippe Bas et Alain Milon, que je tiens à saluer. Ce texte est une étape vers la sortie progressive du confinement. Néanmoins, une question nous paraît essentielle : notre pays est-il préparé au déconfinement ? Dans son discours, le Premier ministre a clairement énoncé un triptyque offensif maintenant très bien connu- protéger, tester, isoler -, qui, selon nous, aurait dû être mis en place bien avant. Derrière ces trois mots, quelle est la réalité ? La première nécessité est de protéger. Le port obligatoire du masque dans les transports en commun constitue certes une avancée, mais il reste une exception dans la sphère publique, où la recommandation continue de l'emporter sur l'obligation. Si nous voulons que les Français soient protégés, ne faudrait-il pas rendre obligatoire le port du masque dans l'ensemble de l'espace public ? Les incohérences successives dans la communication gouvernementale et le changement de doctrine quant au port du masque ont profondément abîmé la confiance des Français en la parole publique. Monsieur le ministre, vous qui faites appel au sens des responsabilités des Français, vous nous expliquiez, voilà quelques semaines, que personne n'avait besoin de porter un masque. Je n'ai pas dit personne ! Aujourd'hui, nous observons un changement de discours du Gouvernement : il devient préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Pour expliquer ce revirement, le Gouvernement a mis en avant un changement de doctrine. Or, depuis le 22 janvier dernier, alors que le virus circulait en Chine, des infectiologues ont signalé la nécessité de mettre un masque pour éviter toute contagion. Au moment où les Français vivent une épreuve inédite, difficile et parfois cruelle, il est important de dénoncer les fausses informations ; néanmoins, avant de prétendre labelliser comme « véridique » telle ou telle information, n'aurait-il pas fallu dire la vérité aux Français concernant la pénurie de masques ?

Or, depuis le 16 mars dernier, le directeur général de l'OMS indique qu'il faut tester le maximum de personnes pour stopper la chaîne de contamination du Covid-19. Les chiffres sont là

sans oublier les équipements de protection pour le personnel habilité à prélever ? Nous avons bien noté l'objectif des 700 000 tests hebdomadaires, mais comment ferez-vous pour l'atteindre, compte tenu des difficultés qui existent dans le déploiement d'une stratégie massive de dépistage ? La troisième nécessité est l'isolement.

Une large palette d'hébergements doit être mise à la disposition des Français qui ne pourront pas s'isoler chez eux, avec toute la logistique qui va avec. Qu'en est-il aujourd'hui ?

sauf pour les personnes entrant sur le territoire. Là encore, ce qui a été annoncé samedi dernier n'était déjà plus d'actualité ce matin. La mesure ne concerne donc que les personnes provenant de l'extérieur de l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni. Royaume-Uni. Nous soutenons la proposition du président Milon consistant à sécuriser, au sein de l'article 6, le périmètre des données de santé. Il est en effet essentiel que les données collectées soient strictement circonscrites et limitées au seul statut virologique du patient. Enfin, dans les circonstances actuelles, nous sommes favorables à la prolongation, prévue à l'article 1, de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet prochain. Cette date, retenue par la commission des lois, nous paraît plus pertinente au regard des incertitudes qui pèsent encore sur les conditions dans lesquelles sera mené le déconfinement.

La sortie de crise repose sur une procédure en quatre étapes : détecter, avec l'appui des médecins traitants et du traçage numérique ; tester, en mobilisant toutes nos capacités isoler et surveiller, dans la limite des libertés individuelles et de la confidentialité des données médicales utilisées. Le Gouvernement a fait le choix de restreindre l'obligation de mise à l'isolement et de quarantaine aux nouveaux arrivants provenant d'un pays extracommunautaire. Dans l'ensemble, le texte qui nous est soumis propose un juste équilibre entre santé publique et libertés individuelles. Nous le savons, l'immunité collective nécessaire pour endiguer la propagation du virus pourra uniquement être atteinte par voie artificielle, c'est-à-dire par vaccination. Pourtant, nous ne pouvons maintenir plus longtemps la France à l'arrêt sans prendre la responsabilité de faire des victimes indirectes, bien plus nombreuses. Il s'agit non pas d'un calcul entre économie et santé, mais d'une équation à multiples inconnues, qui nous oblige à la prudence. En effet, nous ne connaissons pas le nombre réel de personnes asymptomatiques ou paucisymptomatiques ni le degré de contagiosité de ces personnes nous ne connaissons pas non plus la durée d'efficacité de l'immunité des personnes guéries ; enfin, nous ne connaissons pas l'ampleur des dommages que le virus cause à long terme. La distanciation sociale, les gestes barrières, le port du masque : toutes ces mesures élémentaires relèvent de la prévention. Le maillon faible de notre système de santé, trop longtemps

Restons pragmatiques et poursuivons nos efforts pour surmonter cette crise. Les prochaines semaines seront décisives pour les mois à venir ; pour préserver les libertés et la santé du plus grand nombre de Français, le civisme et la responsabilité individuelle de tous

Quel tableau du déconfinement ce texte dessine-t-il ? Une peinture un peu incomplète, parfois même problématique. Commençons par les absences. D'abord, nombre de mesures de déconfinement relèvent du domaine réglementaire. Nous n'aurons donc pas à les examiner, mais, soyons-en certains, la mission de suivi de la commission des lois restera vigilante pour que se poursuive le bon exercice de la fonction de contrôle du Parlement,

Les dispositions du texte relatives à la mise en quarantaine et à l'isolement des personnes entrant sur le territoire national présentent des améliorations significatives par rapport à ce qui était envisagé avant l'avis du Conseil d'État. Le dispositif précédent contenait en effet un risque réel d'atteinte aux libertés constitutionnelles et conventionnellement garanties. Il est heureux que le Gouvernement ait doté le texte de garanties plus solides avant la discussion parlementaire. Parmi celles-ci, nous tenons à relever tout particulièrement le rôle renforcé du juge des libertés et de la détention. Évidemment, pour rendre effectives ces garanties, encore faut-il permettre au juge de remplir son rôle dans des conditions convenables.

; si nous voulons renforcer de nouveau le rôle du juge des libertés dans les circonstances prochaines, il faudra vraiment donner à ce dernier les moyens d'agir dans de bonnes conditions. J'en reviens au projet de loi, car un sujet doit encore être évoqué, celui du système d'information prévu à l'article 6. Nous avons lu les préconisations du comité de scientifiques et l'avis du Conseil d'État ; nous comprenons l'intérêt de procéder à des rassemblements de données pour permettre une lutte plus efficace contre l'épidémie.

données agrégées, même si des précautions sont prises à l'égard des personnes pouvant les consulter, des accidents ou des piratages demeurent possibles. Nous n'écartons pas le principe de la mise en place de ce système,

des mesures dont le pays avait besoin immédiatement, en ajustant ce qui pouvait l'être et en faisant usage de certains raccourcis procéduraux exceptionnels. Toutefois, mon collègue Philippe Mouiller l'a demandé, était-il vraiment impératif de travailler de cette manière cette fois-ci ? N'aurait-il pas été possible, pour le Gouvernement, de mieux anticiper ces travaux dès la semaine dernière, afin d'assurer une bonne information et une préparation correcte des chambres ? Ce texte est naturellement loin de régler toutes les difficultés et toutes les questions qui se posent ; des problèmes entiers demeurent : l'application StopCovid, la responsabilité des élus locaux, en cours de discussion, celle des chefs d'entreprise ou encore les suites des élections municipales ou la tenue des élections consulaires. Nous espérons que les débats porteront sur ces sujets et apporteront une partie des solutions. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains- cela a déjà été dit -réserve son vote à l'issue de la discussion parlementaire. La

d'un plan d'urgence sociale et de suivi des salariés et des personnes en grande difficulté. Je veux donc appeler votre attention sur ces amendements, parce que ceux-ci vous parleront

Soit ! Mais les médecins se sont trouvés dans une situation un peu difficile : d'un côté, il y a le code de la santé publique et, de l'autre, il y a la lettre du ministre. Or, pour l'heure,

médecins l'est aussi, mais à quoi sert un médecin de diagnostic prénatal quand il s'agit d'une IMG pour détresse psychosociale ? Ce n'est pas la question du foetus qui est en cause ; c'est, bien au contraire, la question de l'évaluation de la détresse psychosociale. Par conséquent,

et que, au cas où il ne serait pas adopté au Sénat, vous le déposerez, vous-même, à l'Assemblée nationale. Je vous assure, il est urgent d'agir ; on évoque l'effet qu'aura le confinement sur la prise en charge des maladies chroniques, sur les cancers tardivement dépistés, sur les maladies cardiovasculaires, mais, en matière d'accès aux droits sexuels et reproductifs, nous aurons le même problème. Or nous pouvons l'anticiper et lever aujourd'hui une partie des difficultés. Monsieur